La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur les conclusions du rapport abysses la dernière frontière, à la demande de la mission d'information exploration protection exploitation des fonds marins, quelle stratégie pour la France, je vous rappelle que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes l'orateur disposera alors à son tour du droit de répartis pour une minute, monsieur le Ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura trouvé une place dans l'hémicycle. La parole et tout d'abord à l'orateur de la mission d'information qui a demandé ce départ Monsieur Téva Rohfritsch, rapporteur de la mission d'information pour huit minutes. C'est le rapporteur c'est. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, ce président de la mission d'information, chers collègues, je me réjouis que nous puissions débattent sur les conclusions du rapport que la mission d'information sur l'exploration, l'exploitation et la protection des grands fonds marins adopté le 21 juin dernier le titre que nous avons choisi pour ce rapport bis, la dernière frontière qu'on porte un point d'interrogation, une interpellation bien à propos, tant sont nombreux les défis pour franchir avec Intelligence et discernement, cette barrière de la connaissance. En effet, bien que cela soit difficilement concevable en 2022, il ressort de nos travaux, qu'il nous reste tout. Ou presque, à découvrir des grands fonds marins, ceux-ci s'apparente à bien des égards à une véritable marée incognita et c'est un paradoxe alors que 12 hommes ont foulé le sol lunaire, seuls 4 ont plongé à plus 10000 mètres de profondeur. En conséquence, nous ne connaîtrions selon les plus optimistes, estimation de l'Ifremer que 55 % de la biodiversité de l'océan profond et 2 % de la bathymétrie avec une résolution d'un mètre, cette méconnaissance n'est pas propre à la France qui se situe dans la moyenne des principales puissances maritimes mais la France accuse bien quelques retards sur le plan industriel. En dépit de ses performances reconnues sur le plan de la recherche et de l'innovation, cette situation résulte titre principal des difficultés liées aux grandes profondeurs, mais également il faut le reconnaître, d'un relatif désintérêt de longue date de la part des pouvoirs publics, pourtant les enjeux sont nombreux colossaux, même dans un monde qui va vite et dans la soif de connaissances et de ressources alternatives par insatiable au regard des enjeux de la transition énergétique souvent comparé à nouvelle ruée vers l'or ou encore à la course aux étoiles : l'accès aux grands fonds marins que l'on pense, riche en ressources minérales participe au jeu est en jeu de puissance avec pour compétiteurs, la Chine, la Russie, les États-Unis, la Norvège et de nombreux autres pays en parallèle, il a aussi été démontré, contrairement à ce que nous pensions encore récemment que les abysses abrite une vie abondante disposant de caractéristiques génétiques exceptionnel poursuivi dans ces milieux hostiles ces écosystèmes doivent absolument être préservé, nous ne sommes qu'au stade de la description et non de la compréhension de ces milieux de leurs interactions de leurs fonctions sur ce constat et face à des procédés industriels d'extraction minière sous-marine qui n'ont pas atteint leur maturité, la mission d'information, a estimé qu'il était prématuré d'envisager une exploitation, ceci ne doit pas pour autant nous contraindre à l'immobilisme, nous prenons, au contraire, un soutien accru à la recherche française aux industriels et aux entreprises de service mobilisés sur l'exploration, je suis en effet persuadée que la valorisation, comme la protection de ces milieux fragiles passe par une première étape indispensable de recueil de connaissance, connaître et comprendre pour protéger et préserver telle doivent être nos maîtres mots et je me réjouis, monsieur le Ministre de l'appel à projets, que le gouvernement a lancé le 27 septembre dernier pour 25 millions d'euros dans le cadre du plan France 2030, cette première phase appelle déjà la suivante car les opportunités développement sont nombreuses à titre d'exemple, il faudrait 3500 ans un robot autonome de type à UV pour cartographier l'ensemble de la Z. française, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous annoncer la suite du calendrier pour France 2030 ces enjeux globaux ne doit pas faire oublier la dimension locale et profondément humaine de notre rapport à la mer qui s'apparente à l'intime dans certaines cultures comme chez nous, dans les outre-mer comme chez moi en Polynésie française, la mer, il est considéré comme le 1er garde-manger le trait d'union entre les îles et les peuples, le temple sacré, la voix de l'envol des armes tout simplement le lieu où l'on vit en bord de terre ses dimensions locales et souvent oubliés, comme nous l'ont unanimement signaler les représentants des territoires ultramarins que nous avons auditionnés il est impératif d'associer nos populations nos élus locaux ou ce sera l'échec et le rejet dans nos collectivités du Pacifique, l'impératif culturel, viscéral se joint au respect des lois organiques et de la constitution qui consacre de larges compétences aux collectivités que l'usage local des normes pays non par défiance à la nation, mais par fierté de cette identité particulière en son sein que l'histoire et la géographie en fonder nos territoires d'outre-mer sont bien aux premières loges de tous ces défis, la de française et la 2ème mondial en terme de superficie 97 % de celle-ci est ultramarines quatre 47 % en Polynésie, je ne doute pas, Monsieur le Ministre, que vous trouverez dans ses mots les ressources pour faire naître la concertation mais aussi l'esprit d'initiative y a nuitées Harrouard que l'amour soit grand, dit-on chez nous, dans ce contexte d'enjeux multiples, nous sommes convaincus que la France a un rôle essentiel à jouer sur cet immense deux mais également à l'échelle internationale, elle fut l'une des toutes premières nations à s'intéresser aux grands fonds marins dès les années 60, elle dispose d'un vivier de scientifiques et d'entreprises innovantes de renommée mondiale, la France est un membre historique actif de la IFM qui lui a octroyé 2 contrats d'exploration dans les eaux internationales, ça Marine elle présente sur tous les océans, la France, avec toutes ses composantes ultramarines et donc bien incontournable, c'est une chance pour elle autant qu'une responsabilité que le président de la République a fait sienne nous devons tous ensemble assumer cette responsabilité devant les nations du monde, en particulier celles moins attentive aux impacts de l'émission de l'homme dans ces milieux à Bissau, homme libre, toujours tu à la mer nous disait Baudelaire : la France doit porter au sein de l'AFM une position exigeante quant aux garanties environnementales et aux moyens consacrés à le respect les filles sont passionnants et nous oblige mais ils appellent une forte mobilisation de tous les acteurs concernés, en particulier l'état c'est dans cet esprit de responsabilité que nous avons formulées 20 recommandations il faut notamment monsieur le Ministre, associer davantage le Parlement clarifier la gouvernance aujourd'hui peu lisible et soutenir aussi bien la recherche française que le tissu industriel par une commande publique forte et constante, à ce stade nous recommandations ne porte pas sur l'ouverture de crédits supplémentaires, ni sur l'élaboration d'une énième stratégie mais la confirmation de ce qui a été conçu et annoncé autour de 2 piliers : le pilier civil avec la stratégie nationale d'exploration, d'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins issus de travaux collectifs menée par Jean Louis lever se plier été renforcée par le dixième objectif du plan France 2030 évoquer tantôt le pilier militaire avec la stratégie de maîtrise des fonds marins du ministère des Armées pour le 1er pilier 2 enveloppes normalement, distincte de 300 millions d'euros ont été annoncées, validé par le 1er ministre Jean Castex, il ressort néanmoins de nos auditions que sa mise en oeuvre souffrir et d'un portage politique diffus, trop faible, si telle est le cas, ce serait un échec cuisant pour notre pays, celui de Jules Verne du commandant Cousteau, mais aussi de Pasteur, pourriez-vous nous éclairer Monsieur le Ministre, sur la politique du gouvernement en faveur de la connaissance de nos grands fonds marins avec quels moyens et à quel rythme les 2 budget 300 millions d'euros sont-ils confirmer, quel regard portez-vous sur les 20 recommandations formulées par notre mission au regard des tensions géopolitiques en mer Baltique, vous pouvez-vous aussi nous indiquer si la France dispose de moyens suffisants pour assurer la sécurité de ses infrastructures sous-marines, de communication et d'énergie, de nombreuses questions se posent : Monsieur le Ministre et ce débat, je n'en doute pas, permettra de les éclairer, pour conclure, monsieur le Ministre, chers collègues, je ne pense pas me tromper en soutenant que nous partageons tous ici le souhait classe la France confirme son rang de puissance maritime comme son excellence en matière de recherche et d'industrie sous-marine, nous pouvons relever tous ensemble ce défi de la connaissance avec responsabilité Jules Verne ne s'y est pas trompé en nous invitant à aimer la mer cet immense désert où l'homme n'est jamais seul car il sent frémir la vie à ses côtés, ne s'est donc pas l'immobilisme, mais faisant ensemble la démonstration qu'un modèle vertueux et performant est possible dans le respect des écosystèmes et des fonctions vitales de l'océan, ce modèle doit être porté par la France avec ses outre-mer, merci de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre. Vous souhaitez intervenir. Merci beaucoup monsieur le le président, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices, monsieur le président de cette mission d'information, monsieur le le rapporteur. Je vais être très bref mais je voulais vraiment prendre ce moment pour pouvoir faire un petite introduction d'abord pour vous remercier pour la qualité de de ce rapport, la qualité de ce rapport, dans un contexte en plus ou on connaît très peu de choses sur cette matière et donc je crois que vous avez mené plus d'une soixantaine d'audition 70 pourrait tout à fait précis bien 69, vous avez fait un certain nombre de déplacements, dont un en Norvège, on voit que, dans ce rapport il y a la patte de quelqu'un qui connaît la mère de quelqu'un qui connaît les enjeux de préservation de la biodiversité marine de quelqu'un qui connaît là aussi, les enjeux de valorisation de ce Patrimoine est quelqu'un qui, au fond, mais au coeur de la priorité de la stratégie pour le territoire de la police pour tout le tout le territoire ultramarin et pour la France, la nécessité, hé bien de faire de la merde des enjeux maritimes un enjeu à la fois de lutte contre le changement climatique et en même temps de souveraineté et donc le gouvernement et puis tous ceux qui travaillent sur cette belle politiques ont bien bien pris connaissance des recommandations et nous allons avoir l'occasion à travers les questions des sénateurs et les sénatrices qui vont, qui ne vont pas manquer d'ah d'arriver de peut-être faire trois points de clarification, le 1er c'est qu'il y a un pilote de l'avion, le pilote dans l'avion, c'est le président de la République, puisque c'est une ambition qui est fortement portée, il a eu l'occasion de le rappeler dans les différents sommets le sommet des Nations unies pour les océans à Lisbonne, il a l'occasion de rappeler aussi, dans une belle région que certains nombres de connaissent ici comme le président et l'autre président la la Bretagne de rappeler à quel point la connaissance des fonds marins, la connaissance de l'océan était un enjeu crucial et puis il y a aussi un pilote de l'avion avec une une instance de décision qui est le six, maire, le comité interministériel de la mer où se prennent un certain nombre de décisions ou ces prix d'ailleurs la décision de faire de l'exploration des fonds marins, une priorité et puis il y a une 2ème clarification que vous apportez, et je vous en remercie dans un moment qui n'était pas simple et vous l'avez fait je crois quasiment un peu en avance par rapport à ce qu'a pu porter le gouvernement c'est la clarification sur le fait qu'on devait et que nous n'avions pas nous engager dans la voie de l'exploitation et que ce qui nous guide la stratégie du gouvernement, la stratégie de tous les acteurs, c'est celle d'une meilleure connaissance et celle de l'exploration, celle de la recherche scientifique et donc nous allons avancer dans cette voie là, en incluant bien évidemment tous les territoires, j'y reviendrai, notamment les territoires ultramarins et puis un dernier point de clarification, si je peux me permettent de le faire tout de suite, c'est que l'enveloppe dédiée pour ce magnifique sujet parce que c'est une aventure entreprenariale sinon vêture c'est aussi une aventure industrielle puisque notamment sur la partie militaire, on va devoir là aussi mobiliser un certain nombre de de nos industriels sur le sujet, c'est une enveloppe de 350 millions d'euros, c'est en fait 352 si on compte d'autres petits bouts de crédit qui sont dans quelques ministères, mais aussi une enveloppe qui est forte, c'est un signal politique envoyé pour faire de l'exploration des fonds marins, un sujet prioritaire donc je vous remercie encore à vous aussi d'être présent ce soir pour discuter de ce magnifique sujet parce que c'est un sujet qui a trait à la question de la souveraineté dur l'urgence écologique et d'incapacité au fond aussi à répondre aux grands enjeux pour nos concitoyens et pour les générations qui vont arriver, merci. Merci, monsieur le Ministre, je vous ai permis de de développer complètement même si vous passer un petit peu mais pour la suite, on le sait, à la Rice rester dans le dans le temps. Monsieur Gérard Lahellec pour le groupe CRCE pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Monsieur le président de la mission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme mes collègues, j'ai participé donc avec beaucoup d'intérêt à cette mission d'information sur les fonds marins. J'ai lu attentivement le rapport et je dois dire que je partage l'essentiel des conclusions qui en découlent. En effet, si l'Amazonie, le poumon Vert de notre planète et sollicite à ce type de l'attention du monde au moindre départs de feu nos océans sont sûrement le poumon bleu indispensable à notre avenir, le rôle des océans dans la régulation du réchauffement climatique est indéniable et les abysses en sont peut être la réserve naturellement. Au même titre que nous nous soucions de l'état de nos forêts de nos sols, afin de garantir la qualité, la qualité de notre air, la bonne santé de nos océans doit donc aussi demeurer une de nos préoccupations majeures dans l'intérêt de notre planète et des générations futures, la France a le 2ème espace maritime au monde, il y a donc une responsabilité particulière de ce point de vue-là ne nous comparons pas à ceux qui sauterait les étapes, passez-moi l'expression. En sautant des étapes en confondant vitesse et précipitation et en espérant trouver ici, j'allais dire une nouvelle manne une nouvelle manne énergétique. Une nouvelle manne peut être économique. Peut être une nouvelle manne financière, on sait que l'enjeu est trop important pour jouer à ce jeu là. Alors que le président de la République souhaitait, je le cite, en octobre 2021. Le départ du nerf de cette dernière frontière que représentent les profondeurs maritimes à l'issue de ces missions d'information, nous appelons en vérité ah de la prudence et qu'il nous soit permis qu'il me soit permis ici de souligner que les infléchissements intervenues depuis ses déclarations sont de nature à me permettent d'affirmer ici que monsieur le rapporteur, vous avez vraisemblablement d'ores et déjà peut être été entendus. Pour autant, la fascination. Que constituent ces fonds marins puisqu'on ne les connaît pas. N'empêche pas l'action. Et notre méconnaissance des fonds marins nous éclaire au moins. Sur la nécessité de mieux connaître, je ne citerai pas ici, Paul Valéry et son regard sur le monde actuel, mais il disait déjà en son temps. Que l'avenir serait cognitifs et qu'il y avait besoin de connaître. Et vous l'avez rappelé monsieur le rapporteur, 4 personnes seulement ont observé les fonds marins au delà de 10000 mètres de profondeur, c'est donc 3 fois moins que les personnes ayant foulé la surface de la Lune. Donc la recherche de la meilleure connaissance des abysses et donc une impérieuse nécessité et pour cela, il faudra des moyens techniques mais aussi des moyens humains, les organismes existent, nous les avons d'ailleurs rencontrer, vous les avez rencontrés aussi je pense à l'Ifremer, que je salue au passage à l'institut français de la recherche, donc l'implantation de la mer au CHUM que nous avons rencontré aussi qui ont déjà quelque notoriété au-delà de nos frontières et il sera aussi important d'associer pleinement et je dirais même de confier sûrement le pilotage du suivi de ce sujet, allez, disons-le à nos collègues d'autres Je pense que la mission telle qu'elle a été accomplie constitue par elle-même une invitation en tout cas, permettez-moi de dire ici qu'il s'agit d'un souhait librement donc exprimer alors en tant que Breton. Et peut être avec d'autres protons qui nous regardent ce soir. J'en suis même convaincu. Et depuis les côtes d'Armor auquel je tiens tant monsieur le monsieur le Ministre, je serai également ravi de participer et de lire les résultats à venir de ses études parce qu'il faut continuer à étudier, elles seront indispensables quand je le redis, et j'en termine, s'il est vrai que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans connaissance n'est que démagogie alors. à bon entendeur et merci de votre attention. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. des citations simplement vous dire que, bien évidemment, nous partageons et le gouvernement, le président de la République a eu l'occasion de le rappeler, notamment à à Lisbonne sortait ensuite je le redis ici de devant vous sur la distinction et le fait que. Souhaitons être dans l'exploration et non pas dans l'exploitation, donc je partage votre prudence je partage aussi votre exigence, vous l'avez dit, j'allais dire en creux non vous l'avez dit de manière très claire sur la nécessité d'impliquer nos collègues d'outre-mer, nous le ferons dans le cadre notamment du CNM, elle le Conseil national de la mer et et du littoral parce qu'on va devoir déployer d'ici un an, la stratégie nationale de la mer et littoral qui inclut une partie grand fonds et donc nous le rose, l'occasion de revenir vers vous avec un certain nombre de propositions d'de manière de vous impliquer et donc je crois que le pilote que j'ai évoqué tout à l'heure, il doit être au niveau politique, le président de la République, la première ministre et puis ici, votre serviteur, au secrétariat Data de la mer, mais il doit se faire avec une exigence d'impliquer de co-construire cette stratégie parce que vous êtes à la fois les premiers acteurs et puis ce qui aussi vivent de plein fouet la question du changement climatique partout sur les territoires, et puis nous partageons l'exigence que vous avez évoquée de partager la connaissance, c'est le dernier point que l'on a évoqué lors du comité de pilotage, France 2030 et on a demandé et on va financer des actions de partage de la connaissance de vulgarisation de vulgarisation de communication de ce que nous faisons parce que je crois que c'est comme ça qu'aussi on peut susciter des vocations et renforcer la sensibilisation de nos concitoyens et de tout le monde à la protection des océans et la biodiversité marine. Merci, Monsieur le Ministre, vous souhaitez répliquer chers collègues. la parole est à monsieur Philippe Folliot pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues et tout d'abord je voudrais saluer le président de notre commission Michel qu'et le rapporteur Téva rupture Autriche pour la qualité du travail qu'ils ont su mener et tout ce qu'ils ont su impulser dans le cadre donc de de cette mission si plusieurs milliers d'être s'humains ont franchi l'Everest, le point culminant de notre planète si plusieurs centaines de personnes de plus de 300 personnes sont allés dans l'espace, si douze personnes douze être s'humains ont marché sur la Lune, seule une poignée sont allés au plus profond de la terre, hein, donc sous la mer ah dans les abysses et ceci montre finalement tout l'enjeu est toute l'importance de la marine on Nita puisque si nous connaissons relativement bien la partie la plus superficielle de nos océans, le reste est inconnue, que ça soit la masse d'eau, sachant que la profondeur moyenne est supérieure à 3800 mètres donc au niveau de nos océans et si nous connaissons cette partie supérieure de la masse d'eau, nous ne connaissons pas l'autre partie, celle qui est la plus profonde, ensuite, nous avons un autre enjeu et un autre élément important, c'est celui effectivement par rapport aux fonds marins à proprement parler, au delà de la masse d'eau et et dans ce cadre, je crois qu'il est, il est important de garder le. Paramètres de sagesse qui a été celui que vous nous proposez et que nous vous proposons : Monsieur le Ministre, dans le cadre donc de ce rapport, celui de la prudence, mais prudence ne veut pas dire naïveté parce que, en droit, il y a ceux qui restent ne lisse et reste communiste, c'est-à-dire les biens qui sont communs à à l'humanité et les biens qui sont à à personne et que dans l'absolu, chacun peut s'approprier, il y a une logique qui a été une logique finalement d'appropriation

de 2 millions de kilomètres carrés supplémentaires que nous avons obtenus en termes de capacité de pouvoir maîtriser les, les, les ressources et les possibilités sur sur ces fonds cet homme point et un élément qui est un élément important, mais pour autant, nous devons avoir conscience que les fonds marins, c'est aussi quand même une réalité économique aujourd'hui 32 % du gaz et du pétrole exploités dans le monde de off-Shore donc viennent de sous la mer, je ne vais pas revenir sur les enjeux relatifs au gazoduc, on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, ainsi que par rapport au câble sous-marin avec tous les enjeux qu'il peut y avoir en terme de sécurité et par rapport à tout cela, moi je voudrais. Moins de terminer mon propos, Monsieur le Ministre, attirer votre attention sur un point, un élément : c'est celui de l'avenir du Nautile, il a été décidé trop hâtivement à mon goût de d'arrêter l'exploitation du Nautile à partir de 2028 pour moi, c'est une erreur plus qu'une erreur, c'est une faute pour plusieurs raisons : la première c'est que ce que peut faire un sous-marin, des drônes ne le feront pas de la même façon, ça c'est le 1er point le 2ème point

la France, ça fait partie des 5 nations qui ont cette capacité à pouvoir aller à moins 6000 mètres de profondeur avec des bâtiments habités et le fait de sortir de ce club fermé

perspective d'économies d'un 1000000 d'euros qui serait assez catastrophique par rapport aux enjeux qui sont prégnants à la matière, je vous remercie. Merci, cher collègue, j'ai été très tolérants. Et donc il n'y aura pas de réplique pour monsieur Folliot, mais pour le ministre, il peut y en avoir une, allez-y monsieur mais. Ne confondez pas monsieur Folliot et moi, même si on se connaît, d'autres bancs merci beaucoup monsieur Folliot, monsieur le sénateur et et je. C'est toute votre application sur ce sujet, peut-être pour vous rassurer, on est dans la prudence ce soir et donc vous rassurer pour vous dire qu'il n'y a pas de naïveté de la part de la France, il n'y a pas de naïveté de la part du gouvernement, on a bien conscience que les fonds marins, les grands fonds marins sont aussi un enjeu stratégique et c'est pour ça que, à côté de ces stratégies de recherche de la connaissance de recherche marine nous avons déployé nous développons avec le ministère des Armées, une stratégie de maîtrise des fonds marins pour être en capacité, notamment sur les câbles sous-marins sur la surveillance de notre espace maritime et le rapporteur connaît bien à la fois ces enjeux là et la nécessité d'accélérer et d'amplifier sur les moyens, notamment dans le cas de de la loi de programmation militaire, notre capacité en mer sous sous le la mère aussi a déployé de l'innovation a déployé des moyens de surveillance et puis pour vous répondre très concrètement sur le Nautile, c'est une des possibilités qui sera donnée dans le cadre des financements, France 2030 je prends l'engagement ici devant vous, de regarder ça de manière très précise pour voir si il est possible s'il est souhaitable, et si nous allons nous engager dans la voie de poursuivre, hé bien le financement de cet instrument, comme vous l'avez très bien dit qu'est stratégique et puis je terminerai peut-être. Pour répondre, non pas qu'on en revient toujours à la Bretagne, mais c'était le même sujet que que vous pour oh répondre au au au, un autre sénateur des Côtes d'Armor pour lui dire que il peut avoir accès aux résultats de la campagne de cet été, c'est disponible sur Internet et c'est le bloc de la mission Herman Dieu De pardon n'est pas Dieu Herman De et donc vous pouvez avoir accès à toutes les informations, c'est aussi un des éléments de partage de la connaissance et de la science, merci. Merci, monsieur le Ministre et je redonne 30 secondes s'il le veut à Philippe Folliot. juste Monsieur le Ministre, par rapport aux non--t-il je je rappelle, c'est un 1000000 d'euros, mais simplement il y a une nécessité de prendre plusieurs années pour former les opérateurs du sous-marin et que si on ne prend pas rapidement la décision de le poursuivre poursuivre et et donc il n'y aura pas cette capacité à pouvoir former, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver avec un sous-marin, les opérateurs et je crois que c'est un enjeu important et je terminerai par le fait que si on veut donner cette dimension de rêve pour nos enfants, il faut aussi que celui-ci puisse être incarné et et donc les opérateurs du dont ils font partie aussi de ce rêve. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Stéphane Artano pour le groupe RDSE pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le le ministre ce président de la mission d'information, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a près d'un an, lors de son discours sur le plan de relance, France 2030, le président de la République me déclarer que les fonds marins, je le cite sont un levier extraordinaire pour la compréhension du vivant, il ne faut pas laisser dans l'inconnue, une partie du globe, si plus de 60 et 11 % de la surface de la Terre est couverte par des océans, les grands fonds marins reste très peu connue, selon les scientifiques, 95 % des océans profonds reste encore inexplorés je rappellerai 3 chiffrent à dessein pour se rendre compte de l'ampleur de cette méconnaissance, il est actuellement recensés, environ 250000 espèces vivantes sous-marine, mais selon Jean-Marc Daniel, directeur de département chargé de l'exploration des grands fonds marins Ifremer on pourrait découvrir vraisemblablement entre 1 1000000 et 10 millions de nouvelles espèces hou la la découverte de nouvelles espèces, les fonds marins recellent de nombreuses ressources minières, très convoité, donc comme le cobalt Maghreb manganèse ou le nickel ces métaux entre notamment dans la composition, faut-il le rappeler, des batteries électriques, élément incontournable pour l'avenir de la décarbonation de la production d'énergie et son stockage, il est vrai qu'à l'heure où l'exploration des grands fonds marins s'accélère dans le monde, la France un des pays pionniers, ça a été rappelé de l'exploration des océans doit aussi renforcer ses efforts pour rester dans la course et maîtriser sa souveraineté dans son espace maritime 2ème plus vaste domaine maritime au monde après les États-Unis, et ce grâce à nos outre-mer, notre pays a souvent été présenté comme un défenseur du monde marin, or dans un contexte où toutes les puissances maritimes renforcent leur développement technologique et leurs programmes d'exploration dans les eaux sous leur juridiction comme dans les eaux internationales, d'ailleurs, la problématique de l'exploitation des grands fonds marins refait surface, il faut noter que l'exploitation minière en haute mer constitue pour de nombreuses entreprises privées une opportunité de développement, en particulier dans le secteur industriel comme la production d'engins sous-marins d'avenir cependant cette exploitation inquiète de nombreux scientifiques et ONG, car elle implique évidemment des dégradations irréversibles de notre écosystème et de la biodiversité, avec notamment un effet immédiat sur la chaîne alimentaire océanique, ces craintes sont plus que légitime et on ne peut les écarter d'un revers de la main, c'est pourquoi je l'ai rejoint un compte à leurs revendications de renforcer avant tout notre connaissance des profondeurs, il s'agit d'un préalable indispensable à l'élaboration d'un cadre juridique d'exploitation minière le plus respectueux de l'environnement possible raison d'ailleurs justifié le moratoire qui a été adopté, Monsieur le Ministre, je m'interroge naturellement sur la position du gouvernement sujet vous avez commencé à déflorer le sujet tout à l'heure en introduction décaler la politique que vous souhaitez mettre en oeuvre pour l'exploration et l'exploitation des fonds marins comprendrait que nous soyons un peu perdu parfois entre la déclaration juillet dernier du président de la République lors de la conférence Zuni dans laquelle il appelle à l'élaboration d'un cadre légal pour mettre un coup d'arrêt à l'exploitation minière des fonds en haute mer et ses déclarations précédentes, soutenons la quête d'une extraction minière en eaux profondes. La publication des excellents travaux de la mission d'information sur l'exploration et la protection des fonds marins dont nous débattons aujourd'hui tombe évidemment à pic. Ainsi je souscris à la recommandation de nos collègues visant à temporiser sur une prospection et une exploitation prématurée des ressources minières dans l'attente d'acquérir une connaissance scientifique suffisante sur la question, néanmoins, comme cela a été souligné par le rapport et rappelé tout à l'heure par un orateur cette prudence ne doit pas être synonyme d'immobilisme et nous extraire de la compétition mondiale, à ce titre, l'État doit s'impliquer pleinement dans la structuration d'une base industrielle et technologique souveraine et compétitive au niveau international, ça été rappelé notamment par notre rapporteur, car nous devons garder à l'esprit que d'autres puissances mondiales comme les États-Unis ou la Chine sont moins timorée en la matière, dans tous les cas, le pilotage de la politique à mener sur les abysses au regard du caractère transversal des enjeux méritent de gagner en visibilité, on ne peut donc soutenir la création d'un ministère de la mer de plein exercice, compétent pour établir une stratégie maritime centralisé pour des fonds marins, comme le propose la mission d'information enfin en tant qu'élus ultramarins, j'insiste sur cette recommandation, ainsi que sur celle de renforcer, en particulier les moyens humains et financiers d'Ifremer notamment quelle que soit la position du gouvernement, cette politique doit absolument associer le Parlement et les Outre-mer aux différents stades d'élaboration de pilotage et de suivi, et vous l'avez évoqué, monsieur le ministre, en effet, la question des grands fonds marins ne doit pas être uniquement abordée sous le prisme des avis des instances étatiques et des experts, l'opposition ferme des habitants de Wallis et Futuna, en 2010 et 2012 doit nous servir de leçon, cette décision doit être prise de manière transparente et démocratique, car elle concerne directement l'ensemble des personnes qui résident dans des régions où les modes de vie, l'économie, la culture sont influencés par l'environnement maritime dès lors nous devons établir tous ensemble une stratégie maritime respectueuse de la biodiversité et des écosystèmes, sans quoi elle pourrait susciter la méfiance des territoires et engendrer ainsi déblocage, j'espère, Monsieur le Ministre, que vos éclairages apporteront plus de visibilité, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup monsieur le le le sénateur. Pour répondre d'abord à votre question qui était pas la première, mais qui était celle qui, au fond, qui était centrale guider à la fois les financements, la stratégie, et puis le travail qu'on aura à mener ensemble la la première, c'est de vous rappeler, en effet, la déclaration du président de la République qui a indiqué à Lisbonne qu'il fallait créer le cadre juridique pour stopper les activités menées en en haute mer et ne pas autoriser des activités nouvelles qui mettrait en danger les écosystèmes, comme nous l'avons fait en France pour les aides carburant. Ceci signifie très clairement que, depuis la déclaration du président de la République à Lisbonne, la France s'engage dans sa stratégie dans ses investissements sur uniquement l'enjeu de l'exploration et d'ailleurs c'est ce qui a guidé tous les financements, les 350 millions qui vont devoir être déployée, mais que dans le même temps, et c'est toute, au fond, la bataille que l'on doit mener aussi à l'international, que ce soit dans le cadre du traité Bibi Engie en en bon grand-breton biodiversité Billon nationale juridiction, c'est la protection de la haute mer parce que même si la France ne s'engage pas dans cette voie là, on a conscience, parce qu'on n'est pas naïf que d'autres peuvent le faire et que donc il nous faut, comme dans tous les sujets, comme en tout temps, arriver à convaincre nos autres partenaires ou les autres pays de s'engager dans cette voie là là et donc il faut arriver à codifier les choses qui ne veut pas dire que nous, nous le faisons et c'est pas ce que nous souhaitons faire c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait sur les Audrey carbure sur la montagne dans dans d'autres endroits, on a été je crois en avance et donc ce que nous disons très clairement, c'est qu'il faut que la France soit impliquée aussi dans les instances internationales pour convaincre que pour protéger notre biodiversité pour protéger nos et sans, il nous faut avoir ce cadre strict qui permette au fond, hé bien de ne pas endommager les océans et la biodiversité marine. Merci monsieur le ministre, une réplique non pas de réplique donc la parole est à Madame Micheline Jacques pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, on ne peut naturellement abordé un sujet maritime, sans parler des mer puisque c'est au tour de la France ultramarine que se situe 97 % de sa zone économique exclusive, équivalent à 17 fois sa surface terrestre comme de nombreux collègues n'ont pas manqué de le rappeler, notre pays est donc bien un pays maritime à la lumière de ces chiffres en peine donc à croire que la stratégie maritime française ne soit pas davantage affirmé le rapport de nos collègues, Michel Canevet et Téva Rohfritsch d'une grande richesse est à mon sens un plaidoyer particulièrement nourris en faveur d'une politique maritime ambitieuse qui doit aller au delà des sur jacente pour partir à la conquête des profondeurs marines avec ce débat, et celui qui se tiendra demain sur la stratégie maritime à la demande de la délégation aux outre-mer, on ne peut que se réjouir de la séquence maritime qui s'ouvrent, preuve s'il en fallait de la vigilance particulière du Sénat sur ces questions, la mission d'information formule ainsi de nombreuses préconisations en vue de dessiner l'architecture du pilotage, la stratégie d'exploration des grands fonds marins, elle ne peut en effet se concevoir sans identifier les acteurs qui l'incarneront et la déploieront à cet égard, il va sans dire que j'approuve la nomination de membres au sein du gouvernement en charge de la mer, mais l'exhortation à une politique ambitieuse est aussi le signe que la volonté politique de l'État dans sa continuité d'ailleurs n'est pas à la mesure du potentiel que recèle la mère française, c'est pourquoi je pense que ce n'est pas tant le rang protocolaire du ministre-qui comptent que la volonté au sommet de l'État au sein du gouvernement tout entier, le Parlement devra en outre être pleinement associés en vue de la sécurisation juridique des grands fonds marins que le vide juridique les qui les entourent, fragilise dans le code minier l'imprécision quant à leur exploitation fait encourir un risque et il s'agit de sécuriser ce Patrimoine pour ne pas laisser se développer des initiatives d'autres pays qui pourrait se faire d'ailleurs au détriment des Outre-mer légiférer, c'est protéger le Patrimoine marin son était grippée et, partant, notre souveraineté la mer étant une partie de notre territoire, où la délégation aux outre-mer rouvre ses travaux sur la différenciation territoriale je suis sensible à la place que la mission accorde aux collectivités d'outre-mer dans la coordination de la stratégie pour les fonds marins si elle juge leur exploitation prématuré à ce stade de leur connaissances, elle invite à se placer dans une logique d'anticonstipation la recherche et l'exploration ouvre là aussi des perspectives économiques et scientifiques qui devrait placer les territoires ultramarins au coeur de la politique des grands fonds marins, c'est depuis la terre que l'on conquiert la mer et de ce point de vue les outre-mer constituent des bases avancées géostratégique mais des bases arrières notamment pour la recherche scientifique, pour autant, les représentants des collectivités ultramarines auditionnées ont unanimement déploré l'absence d'information et d'associations à l'élaboration de la stratégie 2021, elle constitue pourtant un enjeu économique, social, éducatif d'intégration régionale qui mérite d'être repensé avec les outre-mer, et pas seulement pour eux, enfin, qu'ils s'emparent pleinement de ce défi une vision maritime ambitieuse, c'est aussi la possibilité pour les territoires ultramarins de renforcer leurs compétences locales tourner leur jeunesse vers de nouveaux métiers, la cartographie et bathymétrie doit offrir une connaissance précise des grands enfants et partager avec les collectivités, en outre, l'approche globale des travaux de nos collègues, tient compte de la place des populations de leur nécessaire adhésion et l'indispensable respect de leur représentation pour assurer le succès, le succès d'une stratégie plus généralement les profondeurs marines de nos zones économiques exclusives 100 doté d'une richesse minérale exceptionnel, que ce soit en la minéralisation hydrothermales les encres hautement cobaltifères ou la présence de nodules des scientifiques relève pas moins de 27 métaux différents, un déplacement à Brest avec la mission était l'occasion de découvrir le travail remarquable de l'Ifremer, dont le rôle central aux côtés des autres instituts le BRGM, le CNRS et le SHOM, pour citer les principaux mérite d'être souligné, ils valent à notre pays de figurer dans le top 10 des grands pays océaniques oui, la recherche doit être soutenu, elle est la clé de la maîtrise des profondeurs et malgré la période troublée qui impose des arbitrages, la recherche stratégique, ne devrait pas faire l'objet de compromis, nous devons également placé l'industrie au coeur de l'ambition pour les grands fonds marins dans cette politique les outre- mer devront trouver une place de 1er plan et bénéficier des fruits du développement des activités autour des profondeurs maritimes qui les entourent, j'en terminerai par un mot sur la coopération en matière maritime, elle est incontournable et se situe au niveau international et pour une bonne intégration des Outre-mer également régionale, je vous remercie.

Merci beaucoup, madame la sénatrice et maire, merci de votre implication aussi sur ce sujet, comme j'ai eu l'occasion de de le rappeler, bien évidemment, à la fois dans la lecture et puis la mise en oeuvre des recommandations de ce rapport, nous avons une attention toute particulière pour les territoires ultramarins pour être très concret à quel niveau les territoires ultramarins les collectivités d'outre-mer vont être impliqué, d'abord parce que cette politique sa stratégie maritime qui intègre la stratégie des grands fonds et porté au plus haut niveau de l'État avec le 6 SIMR ce comité interministériel, il y aura bien évidemment, le ministre des Outre-Mer et bien évidemment, toutes les collectivités qui travaille ensuite dans la déclinaison il y aura le comité le pardon, le Conseil national de la mer et du littoral, qui inclut dedans des élus d'outre-mer des, des, des personnes qui représente, c'est magnifique, territoire et puis ce que je vous propose parce qu'on a besoin aussi d'avoir parfois un peu plus de temps, d'avoir des cadres informelle, il y avait un groupe de concertation qui existe et qui est pilotée par le secrétariat général à la mer et qui, au fond, coordonne administrativement tout ça donc nous allons intégrer tous les élus des Outre-Mer qui le souhaitent, pour travailler avec les ONG et les scientifiques pour hé bien faire entendre la voix des Outre-Mer mer et tout ça servira à nourrir la stratégie nationale mer et littoral qui sera déployée en 2023 et puis nous allons aussi développer, déployer cette planification stratégique des grands fonds marins et donc ça veut dire planification stratégique se mettent en lien aussi avec les stratégies des territoires parce qu'on sait bien que, hé bien les élections ne sont pas toujours au même moment, et donc il y a des stratégies qui sont faites par un territoire et puis la stratégie nationale et puis la stratégie ministérielle et donc cette planification stratégique du territoire français des de la zone maritime française, elle se fera avec cette volonté de porter d'ici 2023, une véritable planification stratégique des grands fonds marins qui se fera, territoire par territoire, avec bien évidemment cette ambition nationale cette implosion pour notre nation. Merci, monsieur le Ministre, chers collègues, pas de réplique. Pas de répit que la parole est à monsieur Joël Guerriau pour le groupe, les indépendants pour cinq minutes merci monsieur le président, Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les Français aiment la mer, mais ils la connaissent mal, disait Jacques Chirac, la surface maritime de la France est, en effet, ça vient d'être appelé 17 fois supérieur à sa surface terrestre, c'est-à-dire à quel point il est difficile d'appréhender la présence française sur tous les océans, c'est vaste espace qu'on tienne un grand potentiel de ressources maritimes parmi celles-ci se trouvent les ressources de nos fonds marins et nous ne connaissons que très peu ses fonds, tout le monde l'a rappelé, il est en effet relativement difficile et coûteux, bien sûr, d'explorer les abysses, surtout lorsque les profondeurs se comptent en milliers de mètres de précieuses ressources minières sont néanmoins susceptibles de s'trouver, nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à ces ressources, en Europe, l'Allemagne et la Norvège sont en train de creuser l'écart, elle reste bien sûr encore très loin derrière les 2 superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Certains pays s'intéresse de près à noter. Notamment dans le Pacifique, pour les ressources qu'qui pourraient contenir mais aussi car nos fonds contiennent des infrastructures stratégiques câble de communication mais aussi pas Line de récents sabotages, souligne le caractère stratégique. Ainsi que la volonté de certains acteurs de les instrumentaliser l'une de nos premières priorités doit être donc l'exploration. Dresser l'état des lieux de nos fonds marins est indispensable pour préserver efficacement notre biodiversité, cela l'est tout autant pour déterminer l'existence de ressources minières, il nous semble à cet égard que la France doit investir suffisamment de la technologie pour mieux contrôler ces espaces maritimes les drôles sont une technologie particulièrement utile à l'exploration sous-marine, il est essentiel que nous puissions la maîtriser. Les recommandations du rapport d'information traduisent la nécessité d'investir ce sujet, notre groupe est bien sûr favorable au renforcement du rôle du Parlement dans le développement de ces projets, il est nécessaire de parvenir à des solutions équilibrées. Pour permettre à la France d'avancer, nous sommes également très favorable au retour. D'un ministère de la mer de plein exercice, cela contribuerait à redonner toute sa place à cette dimension majeure l'histoire démontre amplement que la maîtrise des mer est une nappe est un important facteur de puissance et puis petit paragraphe sur la Bretagne, monsieur le président, mon cher Michel Calvez le mercredi 24 octobre 2019 reste gravé dans ma mémoire avec amertume nous débattions de la loi relative à la délimitation des régions nous défendu ensemble une Bretagne à 5 départements, nous voulions créer un pôle mondial de compétitivité Mer conciliant tous les domaines de l'innovation, de la recherche jusqu'à la construction navale qu'honnêtement la Bretagne à 5 départements, c'était la constitution d'une vraie région maritime avec en façade de grands ports Brest et Nantes Saint-Nazaire la la Bretagne berceau naturel berceau naturel des activités en lien avec la mer et tu ne portes naturel pour conduire une grande politique maritime utiles à l'ensemble de la France à l'heure où l'essentiel du trafic mondial de marchandises s'effectue par voie maritime, nous n'avons pas été entendus et aujourd'hui nous constatons une perte de compétitivité des ports français, avec des besoins d'investissements importants, j'ai bien entendu Monsieur le Ministre, qu'il y aura une coordination nationale il y aura un peu moins de région est plus marqué sur la le maritime, ça serait plus simple, il n'est pas réaliste. De croire qu'avec des moyens limités, la France serait en mesure de rivaliser avec des capacités américaines ou chinoises. Ils restent bien entendu indispensables que notre pays soit en mesure de garantir sa souveraineté sur l'ensemble de ces espaces pour être crédible, tout en tenant compte de nos capacités, la France peut compter sur la conclusion de partenariats avec des avec des puissances qui partage ses intérêts en juin dernier, monsieur le ministre et le ministre des de de nos armées, de la défense. à signer un accord de soutien logistique avec Singapour. Nous nous en réjouissons puisqu'il bénéficiera aux armées de nos 2 pays et nous ne disposons pas de moyens militaires qui nous permettent de contrôler intégralement les vastes étendues de ceux qui sont sous notre juridiction, à l'inverse, Singapour détient d'importants moyens, mais n'a pas l'espace suffisant pour les déployer cela pourrait servir de base à d'autres que partenariat plus globaux qui permettrait donc de protéger notre Patrimoine marin, j'espère que la construction d'un nouveau porte-avions, il y a parfois quelques bruits sur la question, se fera bien comme prévu en renforçant nos coopérations et alliances face à des superpuissances qui ne cessent d'envahir des espaces marins nos partenaires européens disposent en effet de capacité significative la Suède actuellement construire la coque d'une frégate de 7000 tonnes une frégate de 7000 tonnes, c'est ce que c'est, plus que n'importe quel autre frégate que nous ayons en France et nombres de systèmes sur cette régate qui ont été embarqués sont français, les fonds marins seront l'un des prochains enjeux de rivalité entre les États, il faudra bien sûr être en capacité de défendre nos intérêts, il se constituent ses fonds marins d'importantes sources de développement économique, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer et comme je vois que le président regarde mes notes, c'est une étape s'est bien terminé Monsieur le Président, rassurez-vous, j'ai tenu le vrai. Merci, cher collègue. Monsieur le Ministre.

vous avez cité quelqu'un, je cite aussi hein. Un grand breton qui disait sur notre nécessité aussi de renforcer la connaissance de nos concitoyens à la mer, Éric Tabarly, qui disait la mère, c'est ce qu'ont les Français dans le dos quand ils sont à la plage, je crois que depuis on a fait beaucoup de progrès et on essaye de le faire ici en tout cas ce ministère mais il y a un enjeu, là aussi, partout sur le territoire de sensibilisation et de plus grande connaissance je vais essayer de je sais pas vous convainc mais en tout cas vous essuyez à quel point le fait d'avoir un secrétariat d'État placé auprès de la Premier Ministre permet justement de répondre à tous les enjeux que vous avez évoqué puisque étant rattachée à la première ministre, nous avons, j'ai la légitimité d'agir en interministérialité et on voit bien que les enjeux maritimes les enjeux de la mer, c'est à la fois le littoral donc la terre, c'est à la fois les les fonds marins s'à la fois la haute mer, c'est l'économie c'est l'écologique, c'est le défense et le militaire, c'est l'aménagement du territoire et donc je le vois tous les jours avec beaucoup de force, à quel point ça m'évite beaucoup de réunions interministérielles, ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement et puis ça me permet de mobiliser tous les services de l'État pour atteindre cet objectif est bien de faire de la mère de faire de l'océan, un objectif prioritaire. Et donc, avec notamment le secrétaire général à la mer et puis, surtout, la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture, c'est plus de 300 agents c'est six mois que cette direction existe, ça nous permet de déployer cette fonction interministériel de le faire du mieux que nous pouvons, mais je crois, mais beaucoup plus d'efficacité, de cohérence et de convergence et donc sans enjeu, notamment de la maîtrise de des des fonds marins, au fond, fond, reconnaître que la mer est un enjeu de compétition stratégique, hé bien, j'arrive à le faire, nous arrivons à le faire de manière beaucoup plus efficace, parce que justement nous sommes rattachés à la première ministre et donc nous pouvons déployer avec le ministère de la Défense, avec le ce Zarya générale de la défense nationale, une stratégie convergentes coordonnée, cohérente sur l'exploration, la connaissance et en même temps cet enjeu de sécurité, de surveillance et de contrôle de nos espaces maritimes, donc vous le voyez, je sais pas si vous avez convaincu, mais je vous ai démontrer à quel point c'était intéressant et important d'avoir ce rôle interministériel pour les enjeux maritimes. Merci, monsieur le Ministre, pas de réplique, la parole est à monsieur Jacques Fernique, pour le groupe écologiste que Solidarité territoire pour cinq minutes. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la mission de rapporteur, chers collègues, je vais commencer par une citation dont je crois que nous allons finir par la connaître par coeur, vu que ce dossier, le troisième à l'affaire, mais je pense qu'elle le mérite, ouvrons les guillemets, nous devons élaborer un cadre légal pour mettre un coup d'arrêt à l'exploitation minière des fonds en haute mer et ne pas autoriser de nouvelles afin d'éviter qu'mettrait en danger les écosystèmes, ce sont donc les termes exacts par lesquels le président de la République, le pilote de l'avion à définir la ligne française à Lisbonne en juin cette clarté il faut le dire à trancher avec la confusion, les ambiguïtés qui jusqu'ici caractérisé la politique française à l'égard des ressources minérales des fonds marins, défaut de lisibilité dont le rapport de notre mission d'information, a dressé le juste constat : notre mission, a pointé d'ailleurs, je cite, un éclatement de la gouvernance entre divers ministères, dont aucun ne pas rejouer de véritables rôle fédérateur la stratégie française Brouillet dans 3 démarche différente, celle du rapport Lever, qui vient de revoir la stratégie 2015 sur l'exploration et l'exploitation minière qui fut notre rapport de mission l'indique un échec la stratégie militaire, qui travaille à maîtriser tout ce qui se joue de Sensible dans les profondeurs, enfin, on le sait, la stratégie financière, France 2030, qui a fait que 310 millions d'euros spatial et à la mer, les déclarations présidentielles lors de l'annonce de cette stratégie, France 2030, avait des accents très très enthousiaste pour l'eldorado Russell en je cite 84 % des réserves de nos minerais, on comprend donc que la déclaration de Lisbonne, celle que je citais, en ouverture, se positionnant contre l'exploitation minière des océans et en faveur d'un cadre légal international contraignant et surpris, ce qui avait jusqu'ici cru comprendre que l'exploitation industrielle des grands fonds était à terme le cap fixé notre débat d'aujourd'hui et donc particulièrement bienvenu parmi les questions qu'il soulève, Chelsea est centrale, est ce que la déclaration du président de la République à Lisbonne se traduira concrètement par des actes pour changer une donne jusqu'ici particulièrement inquiétante une donne inquiétante si elle devait déboucher sur la voie conduisant à l'extraction minière, alors que ce que je retiens moi comme 3 éléments principaux des auditions de notre mission d'information, d'abord la la méconnaissance considérable, ça a été dit, du fonctionnement des écosystèmes des fonds marins des équilibres fragiles d'absorption du carbone par les océans déstabiliser tout cela pourrait avoir de très graves effets ensuite la grande vulnérabilité des écosystèmes profonds, les impacts ravageurs des expérimentations qui ont été menées dans les années 70 ont ont montré que la restauration de la biodiversité des abysses et terriblement lente enfin 3ème élément une rentabilité économique vraiment pas avéré face à l'extraction terrestre et surtout au potentiel de l'économie circulaire, rien que l'énergie à déployer pour remonter des matériaux, des abysses et et particulièrement rédhibitoire, donc la la première mise à l'épreuve de la déclaration de Lisbonne a été, en juillet, le Conseil de la IFM, sur la perspective d'un code minier on peut regretter que la France n'ait pas saisi ce moment pour être aussi ferme que le président à Lisbonne, certains s'attendaient à ce qu'elle renforce les tenants du moratoire, l'échéance de la règle des 2 ans posées par l'état de Norouz approche déjà de nombreux États s'oppose à l'adoption d'un règlement à horizon, juillet 2023, il préconise plutôt une pause dans les négociations pour avoir le temps d'entamer un travail approfondi qui mène vers un cadre juridique solide et protecteur de la biodiversité marine, que notre pays souhaite gagner du temps dans les négociations qui vont conduire à l'adoption d'un code minier, le président a évoqué la conférence des Nations-Unies sur les océans de 2025 comme étant approprié, il serait raisonnable de continuer à pousser en ce sens cette fameuse règle des 2 ans constitue aussi un flou juridique qui mériteraient une analyse claire bien que la France, je le sais n'interprète pas, c'est très comme une obligation pour le Conseil d'approuver provisoirement de manière automatique toutes demandes déposées à partir de juillet 2023 cette règle constitue une menace à ce jour, en ce qu'elle pourrait permettre l'approbation de licence, monsieur le Ministre ces ambiguïtés qui persistent doivent impérativement être clarifiée pour engager négociations plus à l'avenir, la France, c'est-à-dire tous les services et personne en charge du sujet son pose-t-elle fermement à l'exploitation minière et s'engage-t-elle à interdire l'exploitation minière dans les eaux territoriales françaises d'abord la France confirme-t-elle de façon claire, son opposition à l'adoption du code minier d'ici juillet 2023 et s'assure à ce titre qu'un travail collectif et robuste entrepris à à l'issue du délai de 2 ans, dès juillet 23 la France soutient-elle le principe que toutes les demandes de délivrance de licence provisoire d'exploitation soit fermement rejeté en attendant qu'un cadre réglementaire solide et protecteur des habits soit adopté, enfin, je termine au moment où des problèmes de gouvernance, de transparence, de l'AFM sont mises en lumière : est-il tolérable par exemple que son opaque commission LTC autorise dans une procédure très peu démocratique, peu transparente et absolument pas inclusive la société canadienne TMC d'effectuer des tests dans l'océan pour me remonter 3 3600 tonnes nodules, excusez du peu, de quelle façon, par quel moyen la France oeuvre-t-elle en faveur d'une réforme de la IFM, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre.

important pour la préservation de la biodiversité pour la préservation de la haute mer et en même temps, pour répondre très clairement à votre question, il n'y a pas d'ambiguïté, et il y a une clarté une clarté de dire que la France ne s'engage pas dans la voix et ne souhaite pas l'exploitation la fois la France pardon s'engage dans la voie de l'exploration de la connaissance de la recherche scientifique et Marine et dans le même temps, nous constatons la nécessité de ne pas laisser les eaux laisser la haute mer au fond à la privatisation, à une forme de monopolisation pour des activités qui serait et donc c'est la raison pour laquelle partout dans toutes les instances internationales multilatérales, nous nous battons pour faire reconnaître c'est pour travailler sur un cadre contraignant et pour répondre à votre question, très clairement, aussi sur les actes entre exploration exploitation acte numéro un dans les appels à projets dans France 2030, il n'y a que des projets pour l'exploration aucun explicite sur l'exploitation, deuxièmement, vous l'avez évoqué aussi la France en 2022 a modifié son code minier pour justement pas pouvoir engager ce ce ces ces pardon ses activités cette entreprise d'exploitations donc à la fois la France a dit très clairement uniquement exploration, nous l'avons acté dans le code minier et nous du bâton à l'international, que ce soit, P&G ou au sein de l'AFM pour renforcer et et pour construire ce cadre légal parce que l'AFM et la déclinaison en fait de la conférence de Monte Gobé et c'est le cadre légal en tout cas le cadre que nous n'avons pour l'instant pour discuter. Merci, monsieur le Ministre trente secondes chers collègues. j'aurais aimé entendre la même clarté au au moment des auditions que nous avons menée dans les mois précédents, j'en suis très contente cette clarté, ceci dit sur la réforme de la IFM exprimée par la France, il serait bon de de partager ses demandes nous faire connaître dans quel sens vous souhaitez la réformer et et sur et sur cette fameuse règle des 2 ans et sur son appréciation, il serait bon aussi que votre gouvernement partage son analyse juridique qui serait, si elle était valide rassurante. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Michel Dennemont pour le groupe RDPI pour six minutes. minutes. Le président, c'est le ministre, mes chers collègues. L'évocation de cette mission d'information qui a fourni un travail remarquable, je me suis permis à penser au monde du silence, de Louis Malle en 1956 avec ce 2ème, film de l'histoire des prises de vue sous-marine en couleur, nous vivons de Jacques contexte naïf où le grand public découvre une corne d'abondance qu'il croyait inépuisable, mais entre temps, pas si cet état d'euphorie nous avons déversé durant des décennies, les déchets, les boues d'épuration et des déchets chimiques industriels radioactive ou plastique aujourd'hui la place de l'océan doit être à la mesure de son rôle dans les équilibres climatiques environnementaux et sociaux planétaire, comme l'a répété le président de la République en février dernier lors du sommet de Brest, l'océan et la première victime de ce que nous n'avons pas su faire ou mal fait, je exploitation : pollution, acidification qui l'ont mis en danger, il est donc temps de préserver notre biodiversité et notamment la haute mer, un espace qui commence là où s'arrêtent les zones économiques exclusives des États cet espace nous apprentis à tous, il ne doit toi il ne doit pas être une zone de non-droit, nous ne nions pas que les discussions pour élaborer un texte contraignant visant à sauvegarder cette vaste zone qui couvre près de la moitié de la planète sont difficiles, la ligne d'arrivée est visible, elle est à portée de signatures, mais elle s'est encore évanoui le 26 août dernier à l'issue de 15 jours de tractations difficiles au sein des actions uni parmi les sujets les plus débattus, la répartition des bénéfices possibles issues de l'exploitation des ressources de haute mer ou industries pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques espèrent en découvrir des molécules miraculeuses dans le même temps, nous apprenons qu'une société canadienne testera dans la zone de pluie Burton, espace Icher à notre collègue Philippe Folliot, un système composé d'un prototype de collecteurs de de du le front de la mer, le risque ici, c'est de faire remonter les sédiments et entraîné une perte de la biodiversité et menacé des puits de carbone essentiel et remettre en cause les pêcheries international de ton et d'autres espèces, le temps presse, aussi, le président de la République souhaite mettre en place un cadre au légale pour arrêter l'exploitation minière des grands fonds marins en haute mer, on doit donc continuer à s'activer pour faire entendre cette voix, protection de la biodiversité marine, protection des océans, lutte contre le dérèglement climatique et capture du carbone, nous savons que cette ligne n'est pas partagé, outre certaines grandes puissances économiques, c'est toute une sphère privée qui est engagé dans une course au fond marin. Mais il n'y a aucune honte à défendre la sobriété énergétique, plutôt que de l'épuisement de nos ressources, le réchauffement climatique, et en particulier le phénomène El Nino, entraîné des blanchissement massif des coraux, particulièrement dans l'océan Indien au Japon et dans les Caraïbes en tout. La planète a perdu 14 % de ses coraux entre 2009 et 2018, le rapport de mission de Jean-Louis Levet nous le rappelle l'océan constitue la principale source de protéines pour 3 milliards d'être s'humains et fournir la moitié de l'oxygène que nous respirons, représente l'un des principaux réservoirs de la biodiversité dans le monde, notre voix, notre de voix et donc de préserver cette mise en garde ne doit pas occulter notre besoin de connaissances, la mission d'information, le souligne d'ailleurs très bien six 100 % des fonds marins ont été quant aux graphies par satellite, la résolution obtenue par ce moyen inadapté au fond marin et de l'Ordre du kilomètre, voire de la dizaine de kilomètres, ce qui est évidemment insuffisant pour de l'exploration fine, dit autrement, il n'est pas logique qu'on puisse faire des projets pour atteindre Mars, la Lune ou faire des missions spatiales prometteuse mais qu'on néglige nos fonds marins à l'instant d'émission réalisée par Cousteau qui nous a permis de découvrir la féerie de l'or bleu, nous devons poursuivre nos recherches en direction de cet horizon sans lumière en concis nébuleux ainsi le gouvernement a constitué un comité de pilotage ministériel, celui-ci s'est réuni à plusieurs reprises, la première session s'est tenue sous la présidence des ministres en charge de la mère de l'industrie et de la recherche en février 2022 le fil directeur de ce comité et la mobilisation de crédits publics pas des appels d'offres, encourageant l'exploration des fonds marins en étroite association avec la communauté scientifique, la dynamique est enclenchée, nous devons la poursuivre Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous expliquer le but de ce comité va-t-il être réunis à nouveau pas participer de la volonté de la France d'accroître ses connaissances scientifiques sur les grands fonds marins je vous remercie pour votre attention. Merci, cher collègue. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup monsieur le président, monsieur le sénateur, d'abord je je partage ce que vous avez parfaitement explicitée, sur le fait de retrouver, au fond, le fils de l'aventure maritime susciter des vocations et puis faire naître partout sur nos territoires, notamment à la réunion des futurs scientifiques des futurs chercheurs des explorateurs qui vont contribuer à mieux connaître nous essayons pour répondre très précisément à votre question, vous avez raison, ce qui me permet de peut-être clarifier la gouvernance aussi de ces enjeux de grands fonds marins j'ai réuni avec le ministre de l'industrie, le ministre de la recherche, l'enseignement supérieur, un comité. De pilotage des grands fonds marins il avait comme objectif à la fois de faire le point sur la mission numéro une mission qui a eu lieu à Mayotte et puis surtout de lancer l'appel à projets de 25 millions d'euros sur les grands fonds marins je vais ici explicités quelle était la nature, quelle sera la nature de ce de cet appel à projets de 25 millions d'euros, c'est pour financer des projets de recherche, de développement pour construire des équipements, des drônes, des navires et notamment travailler sur leur et donc, il s'agira avec cet appel à projets de vingt-cinq millions d'euros de développer des sous-systèmes des capteurs des composantes adaptés à ce milieu marin, mais aussi des logiciels et des traitements de données nous avons à l'occasion aussi de ce comité de pilotage de grands fonds marins annoncé un programme d'équipement prioritaire de recherche comme des drônes et quatre missions exploratoires scientifiques sont prévus de cartographie d'analyse de l'activité sismique du volcan de Mayotte d'un drone scientifique et d'un robot d'intervention, vous le voyez, ce comité de pilotage de l'objectif numéro 10 de France 2030 avec un triple objectif : d'abord réunir toutes les parties prenantes, tous les ministères, des ambassadeurs et son nombre de six tous les acteurs de cette belle mission, deuxièmement, faire le point, tirer les leçons de ce qui a été fait depuis déjà quelques années et puis de redire qu'il faut donner à la France, aux chercheurs, aux scientifiques à tous nos organismes de recherche comme le notamment le CNRS ou l'Ifremer, les moyens de faire de la France une puissance scientifique et donc le prochain se réunira au début de l'année prochaine pour continuer à faire le point et continuer à porter cette dynamique, je vous remercie. Merci monsieur le ministre, la parole est à madame Angèle Préville pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour cinq minutes. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la mission, mes chers collègues, l'Humanité a dépassé les limites de la capacité de charge de la planète et s'aventurent toujours plus loin en en territoire non durables, voilà ce que dit aujourd'hui dans le journal Libération Jorgen Randers, professeur émérite de stratégie climatique à Oslo, un des auteurs du fameux rapport Meadows ce rapport intitulé les limites de la croissance publiée en 1972 il y a 50 ans déjà, alors que nous commençons tout juste à agir dressé le constat alarmant de la croissance exponentielle physique dans un monde fini, en effet, la quantité de ressources naturelles utilisées par personne et par an dans le monde, être toujours en croissance et c'est ce que j'appelle la croissance physique de fait 6 des 9 limite planétaire ont déjà été dépassées nous habitons un monde qui se dégrade sans cesse, allons nous refaire les mêmes erreurs dans les abysses, comme nous l'avons fait sur les Terres car une extraction ne peut se faire sans dommage collatéral l'exploitation impacte forcément l'environnement et présente des risques non négligeables pour les être vivants habitants les profondeurs coraux d'eau froide crabe yéti Vert, tu Bicol Anémone transparente, ce sont des écosystèmes uniques plongée dans l'obscurité, où l'on trouve ces espèces endémiques les abysses abrite ainsi une grande diversité biologique que nous ne faisons qu'entrevoir et qui promet de superbes découverte mais notre mode de vie implique une consommation de plus en plus fortes de métaux et de Terres rares et induit une utilisation importante d'appareils numériques de véhicules électriques le le développement indispensable des énergies renouvelables, face au défi énergétique va nécessiter une consommation accrue de ses ressources face à ces 2 enjeux contradictoires, préserver et produire une sensibilisation du grand plus public devient une nécessité afin d'atténuer la pression qui s'exerce sur la recherche de nouveaux gisements et justement les grands fonds océaniques sont riches en ressources minérales et l'état actuel du monde nous montre bien la nécessité d'être plus indépendant puisqu'aujourd'hui la majorité des métaux viennent de Chine, 3 types de minéralisation sont connues à ce jour nodules polymétalliques en hautement cobaltifères et Hama sulfuré toutes ces richesses suscite de plus en plus de convoitise, c'est pourquoi l'autorité internationale des fonds marins doit être confortée avec plus de transparence dans sa gouvernance, mais surtout dans son rôle de contrôle pour la préservation des écosystèmes actuellement seulement 1 % cela a déjà été dit de la haute mer, fait l'objet d'une protection juridique et il faudra aller plus loin car c'est un bien commun sur notre continent, des pays comme la Norvège que nous avons visité avec la mission ont légiféré pour autoriser dans un avenir proche, l'exploitation des grands fonds marins cette exploitation industrielle. Et extraction de minerai sera une nouvelle atteinte au vivant, destruction du milieu habitat iPhone mise en suspension de sédiments et de particules métalliques vibrations provoquant des impacts acoustique perturbations lumineuse puisqu'on est dans des zones de grande obscurité, ce que je viens de mentionner constituera a minima, l'impact des extractions minières, or l'océan produit plus plus de la moitié du du oxygène de l'air, fixe le carbone et constitue d'ailleurs un prodigieux puits de carbone et cela uniquement grâce aux vivants qui s'y trouvent, or le vivant, il est menacé par le réchauffement, vous le savez les pollutions diverses et variées, chimiques, plastiques, sonores qui sont provoqués par l'homme, à titre d'exemple, lorsque nous faisons un prélèvement scientifique en milieu marin, on peut en voir les traces des années plus tard, ce qui est détruit ne se reconstituera pas pas avant des dizaines d'années, car ces écosystèmes se régénère bien moins vite que sur Terre, pour autant, la recherche doit être soutenu et encouragé la France doit se doter, comme le souligne le rapport, d'une filière scientifique marine de 1er plan puisque nous disposons du 2ème domaine maritime mondial, cela est valable pour l'Ifremer et dont il faut accroître les moyens mais aussi pour le CNRS dans lequel 2000 scientifiques travaillent sur le monde marin et bien sûr le SHOM, en effet, nous devons avoir les moyens de garantir notre souveraineté et la sûreté de nos données numériques qui transitent par les câbles sous-marins, sans compter que nos territoires d'outre-mer ne sont parfois reliées que par un câble face aux risques géopolitiques, nous devons maintenir voire même renforcer les capacités françaises d'intervention dans les grands fonds, la découverte des abysses soulève le voile sur un monde fabuleux emblématique de ce qu'est la beauté du monde foisonnante inattendue et pour finir, magnifique, il paraît que chaque prélèvement réel révèle des dizaines d'espèces nouvelles, le seul fait de savoir cela et d'une certaine manière réconfortant : la France sera-t-elle actives à l'international pour oeuvrer à la préservation de la haute mer, en particulier, je remercie le rapporteur et le président pour cette mission très riche et le formidable travail accompli. Monsieur le ministre. Merci beaucoup monsieur le président, madame, madame la sénatrice dans votre intervention, vous avez dit beaucoup de choses sur beaucoup de plans et d'autre chose que j'ai déjà indiqué, donc je vais éviter de me répéter, vu l'heure tardive, pour les débats parlementaires c'est quasiment tous vous dire peut-être sur 3 sujets que vous avez abordés qui sont nouveaux dans le débat qui sont pour moi essentiel, je crois, pour nous, ici aussi, le premier sur la sensibilisation de nos concitoyens, notamment des plus jeunes c'est un enjeu important à la fois pour continuer à avoir un un élan collectif sur une plus grande protection de nos océans, de la biodiversité marine, je le crois aussi pour attirer un certain nombre de jeunes dans les métiers de la mer et de dire que les métiers de la mer, sont parfois méconnus mal connue, font l'objet, au fond d'une vision dépassée et et qu'il y a là une pluralité une pluridisciplinarité, que ce soit géologie océanographie économie aussi l'enjeu entre le littoral et la mer, l'enjeu bien évidemment d'arriver à connecter tout ça avec les nous aux nouveaux enjeux, pardon de câble sous-marin de surveillance de protection et d'autonomie stratégique, et donc la sensibilisation des publics les plus jeunes, en fonction aussi de ce qu'est la réalité des territoires, on ne parle pas de la mer de la même manière dans un en territoire que vous connaissez bien, qui connaît très bien ses enjeux dans un autre, ou l'accès à la mer est quand même beaucoup plus s'éloigner et donc c'est pour cela que dans le cadre de France 2030 nous avons financé une mission en au milieu de l'Atlantique, c'est un tournage qui a été réalisé avec des journalistes, des documentaristes qui justement à pour but de vulgariser ces enjeux de mieux les faire comprendre, pour que chacun comprenne aussi les enjeux de la consommation que l'on fait au quotidien notamment dans tous les outils électriques, électroniques et de dire que dans chacun nos téléphones portables dans chacun de nos objets qui nous permettent parfois de voir des magnifiques images de l'océan en l'espace de 2 clics ou de de suite hé bien ça a un impact sur les océans, ça n'a pas que sur la biodiversité, à un moment donné, ça été chercher ça fait l'objet d'une exploitation et donc il faut qu'on soit particulièrement vigilants pour être sobre pour réduire et pour éviter d'avoir un impact sur la biodiversité marine merci. Merci, monsieur le Ministre, pas la réplique, la parole est à Madame Nassimah Dindar pour le groupe Union centriste pour 4 minutes.

en France et pour la France reste ce soir une grande question, alors même qu'une bonne politique de protection et d'exploitation de notre potentiel maritime pourrait être pour notre nation, une solution mes collègues rapporteurs Michel Calvez devoir aux friches ne s'y trompe pas dans le rapport d'information dont nous débattons ce soir quand il parle de faux départ depuis de nombreuses années, pas le vôtre, puisque je pense que vous prenez un très bon départ, Monsieur le ministre, en vous écoutant, depuis tout à l'heure de faux départ ou de gouvernance éclaté entravant la dynamique nécessaire à une vision politique des fonds marins en France car il est toujours utile de préciser que la France est la 2ème puissance maritime mondial après les États-Unis, on l'a dit avant moi, comme il est toujours utile de préciser et de rappeler que 97,5 97,5 % de notre Z E sont liés aux outre-mer et reste pourtant dans l'ombre des collectivités territoriales, que nous sommes à la Réunion, à Mayotte, la Polynésie de la Nouvelle Calédonie de Saint Pierre et Miquelon ou même de la Guyane, il est toujours utile de rappeler que le potentiel économique et géopolitique de nos îles éparses dans l'India Océanie est important : grâce à la Z E dont dispose la France dans le canal de Mozambique à proximité de l'Afrique, les 20 recommandations émises par mes collègues donne dont un nouvel élan à la stratégie nationale telle que souhaitée par de nombreuses au d'autres autorité auditionnée et ses propositions vont dans le bon sens, je me permettrais seulement d'en souligner 2 principales écosystème à préserver, a dit mon collègue a souligné les autres collègues sur le volet de la préservation, je crois que nous avons beaucoup avancé dans nos îles Eparses, nous avons même sanctuariser les Terres jusqu'à abattre 16000 vaches, les îles Saint-Paul et Amsterdam et il est question aujourd'hui d'abattre les rênes qui peuplent les îles Kerguelen, j'ai donc envie de vous dire ce soir que nous pouvons continuer à gérer de façon durable la faune et la flore de ces régions sont devenir des ayatollahs de l'écologie, et cela vaut pour les fonds marins également car il nous faut allier la présence humaine et la préservation de l'environnement dans nos îles Vierges, j'ai presque envie dire ses vices de ces îles Vierges de l'océan Indien, je parle des îles Eparses, bien évidemment, vous l'aurez compris qui reste et des territoires d'expérimentation particulièrement pertinent, une autre région maritime de la France, à côté de la Bretagne, chers collègues, l'information, donc avec la population environnante, avec les élus, avec les collectivités territoriales reste primordial au coeur d'une mobilisation intelligente et partagée qui faciliterait l'acceptabilité sociale des populations impacté aussi nombreux sont les élus qui demandent une coordination entre, par exemple, la Réunion et Mayotte sur une vision partagée des fonds marins en matière environnementale, comme en matière économique et au-delà, au niveau de la quand on parle de la CEI, je crois qu'il nous faut aussi quand on n'aborde ce sujet abordé, celui de la coopération régionale avec les pays voisins, les pays de la CEI, avec également la grande île qui est Madagascar s'agissant des énergies marines, un centre de recherche existe aujourd'hui à la Réunion, les travaux sont menés par l'Ifremer, l'IRD, mais quel partage pour assurer l'implication des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et je pense également aux communes littorales qui sont nombreuses sur nos îles en clair, vous l'aurez compris les ressources de l'océan profond leur utilisation durable au service d'une prospérité commune ainsi que l'implication de toute partie prenante dans les choix éventuel en matière d'exploration ou d'exploitation des grands fonds marins ne doit pas se décider en vase clos, mais de manière concertée élargie, je pense que la France, il prend vraiment vraiment le bon chemin et principalement au niveau des recherches en lien avec l'ensemble des outre-mer mais aussi les pays limitrophes, je pense par exemple à l'Australie dans le domaine des géosciences marines le 2ème point sur lequel je souhaiterais attirer l'attention du ministre et ce livre de la flotte outre-mer et la dotation en drônes sous-marins, mais vous avez quasiment répondu à la question, le rapport note la nécessité d'accord il y a des patrouilles à grands font des patrouilles aux grands fonds en lien avec l'industrie française là dessus, vous nous avez aussi livré que d'ici 2025 nous aurons six patrouilleurs dont 2 à la Réunion et je m'en réjouis, je pense que je peux et que nous pouvons compter sur votre implication en tous les cas au ministère de la mer, les outre-mer attendent beaucoup de votre travail en lien avec nous-mêmes, on vous remercions. Monsieur le Ministre. vous avez là aussi dit beaucoup de de. 2 choses à la fois sur la stratégie, puis la nécessité d'impliquer, c'est à la fois la vision et puis la méthode d'abord vous dire et là, nous devons reconnaître, en tout cas le gouvernement doit reconnaître qu'on doit aller beaucoup plus loin sur la stratégie que vous avez évoqué un Océanie. C'est bien comme ça que nous devons dire on a. En fait, depuis 5 ans, un travail je crois approfondie en lien avec les différentes collectivités locales sur la stratégie indo-Pacifique, je crois que nous devons entamer et faire le même travail sur la stratégie, hein, d'Océanie en lien, bien évidemment, avec tous les autres territoires tous nos 7 pays et donc je vous invite, là aussi à travailler avec nous, en tout cas, nous nous y impliqueront pour faire en sorte de développer une stratégie et une vision ensuite, vous avez parlé au fond de la force des territoires pour réfléchir à tous ces enjeux ces enjeux de valorisation ces enjeux suis de souveraineté alimentaire puisque quand vous êtes à la Réunion, l'océan est aussi un enjeu fondamental pour l'autonomie alimentaire et donc la nécessité la capacité aussi aussi à moderniser la flotte, je sais que c'est quelque chose que vous portez, que nous allons continuer de porter avec notamment le ministre des Outre-Mer et donc l'invitation que je vous fais la proposition, c'est dans le cadre de ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur la planification des grands fonds marins hé bien de puiser dans la force de ces territoires dans les spécificités et sur votre connaissance aussi de cet été. Passe pour à la fois travailler sur la valorisation, sur la protection sur la parfois sanctuarisation et puis sur la définition d'une coopération régionale, vous parliez de le on peut parler du Mozambique, on peut parler bien évidemment des États de la et donc on va entamer ce travail dans le cadre aussi du Conseil national de la mer et du littoral on va aboutir de manière je crois raisonnable, c'est-à-dire d'ici l'été 2023 assez stratégique qui se basera sur la force des territoires comme celui de la Réunion, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à Madame Muriel Jourda pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, monsieur le président de la mission d'information, monsieur le rapporteur, mes premiers mots seront bien évidemment pour notre collègue Téva Rohfritsch qui a été rapporteur de ce travail sur une meilleure maîtrise des fonds marins fonds marins dont l'importance n'est plus à démontrer, je crois que les événements récents sur Nord Stream, nous rappelle que les fonds marins, c'est le lieu du transport des hydrocarbures, c'est aussi le lieu où 98 des échanges numériques et des informations numériques circulent et puis c'est aussi le lieu où peuvent se trouver éliminerait les métaux dont nous avons besoin aujourd'hui dans notre industrie et notamment c'est évidemment sur ce sujet que notre rapport s'est attardé et c'est aussi sur ce sujet que je m'attarderai cette question particulière évidemment se heurte à plusieurs obstacles qui ont été tous révélés par ce ce rapport d'information : le premier, bien sûr, c'est celui de la connaissance, la biodiversité n'est connu qu'à hauteur de 5 % dans ses fonds marins et si cela ne doit pas être un obstacle total à leur exploitation, il faut être évidemment vigilants et nous ne pouvons pas exploiter sans mieux connaître cette biodiversité, nous ne pouvons pas non plus exploiter sans mieux connaître ces fonds eux-mêmes les connaissances bathymétrie que porte sur 2 à 5 % du plancher océanique et à la vitesse à laquelle nous allons hé bien il nous faudrait 3500 3500 ans pour les connaître, totalement, il est donc nécessaire de se doter des moyens suffisants de se doter des moyens suffisants, certains ont été très largement précisés par mes prédécesseurs et je n'y reviens pas mais il s'agit bien sûr des moyens à nos organismes publics, je pense à Ifremer au CNRS au bien sûr au BRGM Leader également mais il s'agit également de nos entreprises privées qui ont un rôle à jouer, qui sont nombreuses mais qui manque un peu de Leadership et qui manque surtout de visibilité politique, il faut le dire, j'ai bien entendu Monsieur le Ministre, que vous indiquer à quel point le président de la République était impliqué, mais notre rapport a révélé qu'il n'y avait pas moins de 8 ministères qui était en charge de ces stratégies 8 ministères, dont aucun, à un véritable Leadership en tout cas pas le ministère de la mer, malheureusement, nous l'aurions souhaité, nous avons à côté de ses ministères, le secrétariat général de la mer, effectivement, et vous nous indiqueraient en quoi la nomination de Didier Lallement est un signe positif pour cette stratégie maritime, mais je devrais dire pour ces stratégies maritime, car en réalité cohabitent plusieurs stratégies, ce qui a été aussi révélé par le rapport, bien sûr, le plan d'investissement France 2030, mais également les 6 maires les comité interministériel de la mer et la stratégie des fonds marins également du ministère des Armées dont on a eu quelques difficultés à comprendre comment il s'interpénétrer, de la même façon qu'on a eu quelques difficultés à comprendre si les financements se cumulaient ne se cumulait pas mais nous, vous nous avez donné un chiffre, un chiffre tout à l'heure, et au-delà de cette volonté politique, mais cela s'inscrit aussi dans la volonté politique, il a été rappelé que 97 % de notre zone économique exclusive, se situe dans les territoires ultramarins et les auditions auxquelles nous avons procédé des élus ultramarins ont toutes révélé à quel point ils ont eu le sentiment, et ce n'était pas qu'un sentiment, à vrai dire à quel pourrait, ils n'ont pas été concertés en aucune façon sur ce qui se passait sur leur territoire et alors que, on l'a indiqué tout à l'heure, culturellement, hé bien, la mer peut confiner au sacré dans certains territoires, il ne paraît pas envisageable de travailler sans eux, mais je crois que vous l'avez parfaitement saisi monsieur le Ministre, voilà donc quels sont les obstacles et quels sont les enjeux et ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas de trouver au fond de la mer des minerais dont nous manquerions sur terre car aussi le rapport a révélé que plus nous avons besoin des minerais et plus nous en trouvons sur terre, la situation n'est pas celle-là, l'enjeu est véritablement celui de la souveraineté sur des territoires et dans des domaines où nos compétiteurs sont nombreux et sont agressifs. Il ne suffit pas de devenir une zone économique exclusive de 11 millions de km2, encore faut-il avoir la volonté de refaire de la France une grande puissance maritime et je crois que nous avons tous les atouts pour cela je vous remercie. Monsieur le Ministre. madame la la sénatrice merci beaucoup au de votre intervention, qui me permet de de clarifier un certain nombre de de choses, notamment sur la question de la la gouvernance et je souscris pleinement à vos propos sur la nécessité, au fond, de faire de la France, de continuer à faire de la France une puissance maritime qui ne s'arrête pas simplement à l'enjeu de l'espace de la délimitation qui est d'abord un enjeu aussi de puissance économique de puissance militaire et de puissance scientifique, comme je l'ai rappelé. Le cadre est au fond la gouvernance, elle est très clair : je vais essayer ici de l'expliciter, il y a la mer, c'est un espace et donc, étant donné que c'est un espace il y a plusieurs activités qui s'y joue et donc il y a plusieurs secteurs et donc il y a plusieurs ministères et c'est la raison pour laquelle nous avons avancé ou en tout cas nous avons déterminé que la meilleure manière de prendre en compte cette interministérialité de de la mer et de faire des enjeux maritimes un enjeu écologique un enjeu stratégique est aussi un enjeu de souveraineté, c'était de le placer auprès de la première ministre et donc il y a le 6 maires qui est un cadre politique, le comité interministériel de la mer qui est présidé par la première mise où se font les grandes orientations de la politique de la mer, ensuite il y a une déclinaison politique c'est votre serviteur, le secrétaire d'État à la mer, qui coordonne politiquement tout ce qui se passe sur la mer, c'est ce qu'on devra faire sur la planification maritime pour les énergies marines renouvelables qu'on doit faire en lien avec bien évidemment le ministère des Armées qu'on doit faire en en lien avec le monde de la pêche et donc sur les enjeux que vous évoquiez, dans le cas de la stratégie il y a une instance qui s'appelle le Conseil national de la mer et du littoral qui, au fond, le parlement de la mer, qui regroupe des parlementaires qui regroupe des usagers qui regroupe des associations et qui là aussi est placée sous l'autorité du secrétaire d'état de la mer et qui a la comme objectif de faire cette coordination et puis il y a à côté, le secrétariat général de la mer qui a fait la coordination administrative administrative pas l'animation politique pas l'impulsion politique et donc, vous voyez, c'est clair, il y a le 6 il y a le secrétaire d'État à la mer, et il y a, pour la partie administrative et la déclinaison partout sur les territoires, en lien avec les préfets et les préfets maritimes le secrétaire j'ai général à la mer, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, la parole, il y a pas de réplique si. Madame Jourdain. Merci monsieur le président, mon propos sera brève, je ne suis pas sûr que vos explications apporté beaucoup de clarté, elles ont en tous cas, démontrer que, il y a beaucoup d'acteurs et qu'on on peine à comprendre, malheureusement, quel est leur articulation réel. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, comme de nombreux orateurs précédents l'ont mentionné les océans présentent des potentiels inégalée dans le domaine nutritionnel pharmacologique et que énergétique minier, certains s'emploient à dire que la vie serait issu des océans et qu'aujourd'hui notre survie en dépendrait pourvu que nous sachions exploiter ses ressources de façon raisonnée, ils font aussi l'objet d'enjeux stratégiques et géopolitiques et les conflits terrestre trouvent désormais leur prolongation dans les fonds marins, le rapport qui sert de base au débat de ce soir, insistent sur la nécessité d'une cohérence dans la stratégie et d'une coordination des actions, mais au-delà de la gouvernance, se pose la question de savoir si la France a l'ambition de devenir une grande nation maritime : elle devra comme le mentionne Christian Bûcher s'affranchir de son passé, qui constituait à vouloir desserrer la mâchoire de fer de Charles-Quint et à se tourner vers l'Est, donc vers la terre, l'Exposition Miroirs du monde que l'on peut admirer en ce moment au Musée du Luxembourg, témoigne que la connaissance et la puissance ont dépendu de la maîtrise des maires et de l'organisation des circuits logistiques, comme l'ont fait les Portugais, les Hollandais, les Anglais et aujourd'hui les Chinois affirmait une vocation maritime 7 impulser une identité maritime qui passe par la sensibilisation, l'éducation, la vulgarisation scientifique et technique, la constitution d'un réseau de formation et de recherche, la création d'un pôle d'excellence permettant de structurer une filière industrielle dont l'amorçage ne pourra être effectué, comme le souligne le rapport, dans un 1er temps que par la commande publique, je voudrais souligner les efforts des villes et des régions qui aujourd'hui en France ont lancé de nombreuses initiatives ainsi à Cherbourg, de l'autre côté du du Couesnon en Normandie, qui a la 5 départements, la Cité de la mer qui vient d'être élu monument préféré des Français 2022 accueille en cette fin de semaine, ainsi que l'événementiel dénommé grands océans et cela organisé par Sciences et Avenir et et Les Échos Monsieur le ministre, au moment où la récente nomination du secrétaire général de la mer nous interroge : quelle est votre feuille de route, quelles seront les prochaines actions que vous impulseur pour structurer une véritable filière océaniques sur le plan international, l'exploration et l'exploitation des fonds marins prennent l'allure d'une ruée vers l'or bleu, et cela au détriment de la préservation de l'environnement ainsi au-delà des recommandations du rapport, le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat insiste sur la nécessité de soutenir une initiative diplomatique visant à promouvoir au niveau international, un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, n'excluant pas la possibilité d'intervention pour l'exploration qui devront être néanmoins codifié afin de ne pas détruire les écosystèmes de mettre en place des sanctuaires des profondeurs afin de délimiter des zones qui seraient totalement protégé et qui pourraient être reliées entre elles par des corridors biologiques sous-marin, il est à noter que cette proposition figure dans l'étude, les grands fonds marins quel choix stratégique pour l'avenir de l'humanité, réalisée par la fondation de la mer en 2022, et enfin de refondre complètement l'autorité internationale des fonds marins et notamment réviser son mode de financement basé actuellement sur une taxe perçue sur l'exploitation qui positionne de ce fait, l'autorité dans une situation ambigu cette refonte doit aussi permettre à l'autorité de contrôler et de sanctionner les pays et les acteurs qui contreviendraient aux obligations de protection de la biodiversité de la biodiversité, alors Monsieur le ministre, le gouvernement partage-t-il l'analyse de refonder l'AFM son mode de financement et de lui donner un pouvoir de contrôle et de sanction. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur merci de. Toutes ces questions très vaste, qui vont des objectifs politiques jusqu'à la question de l'AFM très rapidement et le plus concrètement possible, d'abord, l'objectif de ce secrétariat d'État, la feuille de route qui avait été donné, tourne autour de 3 objectifs : le 1er, la protection des océans et de la biodiversité marine à la fois sur le territoire mais aussi à l'international, c'est tout l'objet de ce que l'on porte aussi dans le cadre de Bibiane J. deuxièmement c'est développer l'économie maritime partout sur nos territoires lancé la décarbonation de ce secteur, notamment les ports et les navires et soutenir notre modèle de pêche qu'un modèle de pêche très diverses, que ça va de la Méditerranée jusqu'à en à la manche et puis le 3ème enjeu de 3ème objectif c'est de planifier de lancer cette grande exercice de planification de l'espace maritime parce qu'on le voit bien, la mer est un objet au fond où se multiplient les usages, où il y a une densification et une multiplication et entre les énergies marines renouvelables entre les pêcheurs ou encore dans les activités plutôt touristique, il y a besoin d'avoir cette planification et donc sur le 2ème point le point que vous m'avez interrogé sur la planification et la sanctuarisation pardon c'est cet exercice de planification qui va nous permettre là de répondre à l'objectif qui a été proposé par la fondation de la mer de la sanctuarisation et dans la stratégie nationale de biodiversité, nous pouvons aller vers sa sanctuarisation j'y suis favorable, le gouvernement est favorable à avancer aura besoin de ce cadre de planification en lien avec les territoires, et puis sur le dernier point, le troisième qui est celui de l'AFM, oui, nous sommes favorables à une réforme du financement de l'AFM, nous sommes favorables à au fond adapter l'organisation, le cadre de l'AFM aux nouveaux enjeux et une nouvelle demande à la réalité qui est celui, hé bien de protéger les fonds marins, d'avoir un cadre international qui permettent bien de protéger nos océans et donc nous allons avancer, nous aurons besoin des débats parlementaires pour continuer d'avancer, mais je sais que vous y êtes prêts comme le rapporteur comme les différentes orateurs qui étaient ici avant vous, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, pas de réplique, la parole est à monsieur François Bonhomme pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur rapporteur, mes chers collègues, d'abord je veux saluer ici l'initiative du groupe R des pieds et l'organisation de ce débat qui nous permet effectivement de mettre en exergue la situation notre pays du point de vue maritime l'espace maritime de la France dans les domaines économique mais aussi militaire est un élément constitutif fort de notre capacité d'influence et plus largement de sa puissance, cette mission d'information, nous rappelle fort à propos que notre zone économique exclusive et source d'immenses richesses qu'il nous faut protéger. Protéger pour une raison économique puisque la quasi-totalité de nos échanges transitent par des voies maritimes et la totalité ou presque de nos données internet passe par des câbles sous-marins dont nous prenons conscience depuis quelques temps, combien notre sécurité en dépend Interhome PC Flux et notre vie individuelle et collective, en sera complètement bouleversée et désorganisé cet impératif mettent en exergue le rôle 1er de protection de sécurisation notre Marine nationale que je tiens ici à saluer de manière plus générale approches maritimes de notre puissance et donc essentiel pour des raisons multiples, c'est pourquoi les orientations stratégiques et les capacités de le respecter sont partiellement importante pour peu que nous voulions conserver une capacité de puissance à l'achat de la planète ou tout au moins conforté notre rôle, notre position de puissance régionale de 1er plan, car ces dernières années un certain nombre de signes nous laissent penser que notre zone et Florence a eu tendance à se réduire au regard de d'autres grandes puissances maritimes, c'est d'autant plus dommageable que nous disposons de ressources considérables, je pense bien évidemment aux grands fonds marins certes ils ont figuré dans le plan d'investissement France 2030, or cette mission d'information, nous rappelle combien les enjeux ont été parfois insuffisamment partagée pourquoi ainsi se limiter à quelques experts sous la houlette de l'État pour fixer les grandes orientations, les moyens adéquats, nous rapportons bien souligner combien nous avions besoin d'un petit d'un pilotage clair et élargi, c'est pourquoi, par exemple la désignation d'un délégué interministériel le fond marin en charge d'animer la politique des fonds marins, de coordonner l'action des différents ministères et les acteurs scientifiques est véritablement nécessaire, de même le rapporteur appelle de ses voeux à juste titre la création d'un ministère de la mer de peine exercice pour mettre à l'oeuvre, la politique maritime française, à commencer par les grands fonds marins mais aussi la pêche et l'aquaculture, enfin, pourquoi ne pas impliquer le parlement en désignant présentant de chaque assemblée au sein de du comité de pilotage de la stratégie il y a et y associer les délégations parlementaires aux outre-mer ainsi que les exécutifs ultramarins, De l'ensemble des connaissances préalables avant toute décision de prospection et d'exploitation des ressources minières des fonds marins, elle constitue une option sans nul doute stratégiques mais c'est à bon droit que le rapporteur, ont indiqué combien nous avons besoin de connaissances scientifiques approfondies qui font aujourd'hui parfois défaut sur les grands fonds et leur écosystème alors Monsieur le Ministre, pour éviter toute procrastination, faites en sorte d'écouter le Sénat au moment où tant d'autres puissances maritimes voit de manière de moins en moins voilées ces espaces, nous avons des échos de ce qui se passe dans le Pacifique, ils ne peuvent que nous inquiéter, à cet égard, ou l'implication des États-Unis où les manoeuvres de la Chine sont de moins en moins feutrés, il est véritablement temps de réagir, ce travail d'approfondissement de nos connaissances et d'élargissement des partenariats avec les parties prenantes qui soient les chercheurs, associations, élus ou entreprise est véritablement une étape préalable avant de considérer l'opportunité de poursuivre ou non l'objectif d'une exploration en vue d'une exploitation industrielle de nos fonds marins voilà monsieur Ministre les conditions et l'étape indispensable pour donner, j'espère un nouveau départ à la stratégie nationale pour les grands fonds marins. Monsieur le Ministre. Ma présence ici et le débat qu'on nous avons eu, je crois que vous êtes le dernier orateur qui a un débat riche montre à quel point le gouvernement non seulement écoute mais va faire sienne, un certain nombre de propositions, je l'ai dit tout à l'heure, notamment sur l'implication des élus, des élus des territoires ultramarins sur cette nécessité, comme vous l'avez évoqué d'avoir une planification stratégique, notamment avec des objectifs de sanctuarisation ou encore de renforcer l'interministérialité de renforcer, hé bien la cohérence, la convergence des différentes stratégies et donc nous allons vous écouter, nous avons écouté sur par exemple l'enjeu de mieux prendre en contre, ce qui a été dit et ce qui est dit par les parlementaires, c'est pour ça que j'ai relancé dès la semaine dernière le Conseil national de la mer et du littoral, j'insiste, parce que c'est le Parlement, vous avez évoqué tout à l'heure, tous les acteurs, c'est là où se réunissent tous les acteurs, c'est là ont défini la stratégie, c'est là, on fait de l'évaluation, c'est là où se place la concertation, alors peut-être qu'il n'est pas assez connu, en tout cas, il est très utile, c'est, il me semble en plus quelque chose qui a été porté au moment du Grenelle de la mer par tous les acteurs, et donc je veux vraiment en faire le lieu où tous les acteurs se rassemblent discute et surtout avance et co-construite et puis au Parlement, je crois que, ici, au Sénat, le fait que vous avez ce débat qu'on continuera à avoir ce débat, je me tiens à votre disposition pour continuer continuer d'avancer à la fois sur les investissements, travailler sur la décommunisation, territoire par territoire et puis travailler sur les moyens que l'on doit se donner dans le cadre notamment du PLF pour le CNRS pour l'Ifremer pour l'IRD ou encore pour la flotte océanographique française nous avons et nous allons vous écouter sur l'enjeu au fond d'avoir une une personne qui continue, pas simplement de coordonner mais d'être dans la déclinaison et dans l'écriture, territoire par territoire de ce qui est fait et c'est pour ça que j'ai proposé la création au sein de mon ministère de ce poste de coordinateur de la planification des grands fonds marins qui fera ce travail avec tous les ministères et qui aura pour notamment au rôle principal ou en tout cas pour une démission principal d'écouter ce que dit par le manque d'écouter ce que dit le Sénat et ensuite de le décliner en actions très concrètes, je vous remercie,

Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, d'abord, merci beaucoup pour s'érige essence merci de me donner la possibilité de donner la possibilité à ceux qui nous regardent de pouvoir échanger, discuter, avancer sur cet enjeu passionnant, qui est celui des abysses et des grands fonds marins comme vous l'avez dit les mers et les océans couvrent 71 % de la planète et la grande majorité sont des nommés les grands fonds avec une profondeur entre 200 et 6000 mètres et couvre 65 % du globe, vous le savez la France de par son histoire, de par sa géographie et ses territoires ultramarins est une grande puissance maritime et l'objectif du président de la République et de la feuille de route qui m'a été confiée par la première ministre et de tout faire pour protéger nos espions pour valoriser nos espaces maritimes et de faire de la France une puissance du XXIe siècle, une puissance maritime qui a des actions exemplaires sur son territoire mais aussi à l'international : être une puissance maritime, mesdames et messieurs les sénateurs, ce n'est pas uniquement être une puissance militaire, ce n'est pas une uniquement être une puissance économique, c'est, je le crois profondément et on l'a vu ici et votre rapport l'a parfaitement montrée c'était une puissance scientifique et donc se donner les moyens d'avoir une stratégie pour la recherche marine car comme vous avez pu le voir et le décrire parfaitement durant nos travaux, la connaissance des grands fonds marins et la condition indispensable pour en mesurer. Tous leurs effets pour mesurer ce qu'il recouvre les valoriser mesuré la fragilité et une fine et les protéger, alors nous avons un comité interministériel de la mer, en janvier 2021, celui-ci a fait de l'exploration scientifique des grands fonds marins sa priorité et comme vous l'avez dit, nous n'en connaissons qu'une infime part ils sont moins connus que l'espace et donc nous avons posé ici un 1er cadre et ce comité interministériel de la mer s'inscrit dans une architecture dans une gouvernance et je c'est ici qu'elle a pu faire l'objet d'un certain nombre de questions qui est pour nous très clair : il y a la première ministre il y a le secrétaire d'État à la mer et puis ensuite il y a une coordination que nous faisons, que je fais en lien avec le secrétaire général de la mer, c'est d'ailleurs la même chose sur les enjeux, défense, nous avons un ministre de la Défense, un secrétariat général de la défense nationale, c'est la même chose sur l'Europe, nous avons un Ministre délégué à l'Europe et puis nous avons un secrétaire général aux affaires européennes qui permet de faire cette coordination qui permet de prendre en compte toute l'interministérialité de ces enjeux, et donc c'est prier sa priorité, pardon, je souhaite qu'elle soit mise en oeuvre dans le cadre du parlement de la mer que nous avons qui est le Conseil national de la mer et des littoraux qui, au fond, notre instance de concertation principal qui réunit les usagers de la mer, les ONG, les élus de tous les territoires et les services de l'État, c'est dans cette instance que sera discuté la stratégie nationale pour la mer et lutte orale que nous aurons à construire d'ici 2023 c'est dans cette instance, que nous allons porter les priorités sur les grands fonds marins que nous allons décliner les investissements et que nous allons prendre en compte les spécificités des territoires et pour répondre à votre deuxième recommandation, monsieur le rapporteur je nommerai une personne qui s'occupera de ce pilotage des grands fonds marins qui fera le lien entre l'aspect financier, France 2030 et la planification que nous aurons à établir partout sur ces territoires, c'est cette gouvernance je le crois, qui nous permettra de concerter de faire mieux, de décider et de financer des priorités sur les grands fonds marins qui répondent à tous les objectifs que vous avez définie et puis nous aurons et c'était une des recommandations aussi de vos rapports d'augmenter d'amplifier notre soutien à notre capacité de recherche je pense ici au CNRS à l'Ifremer et à lire des et nous aurons à mobiliser toutes les forces de la recherche française, pour atteindre un double objectif : la préservation de l'océan et l'exploration des grands fonds, vous l'aurez compris ce sujet est porté au plus haut niveau par le président de la République dans le cadre de France 2030 et par la première ministre avec ce comité interministériel de la mer et une coordination qui se fera au niveau de mon ministère, nous devons concentrer et vous l'avez dit, vous avez été plusieurs à l'évoquer toute notre attention, tous nos financements sur l'exploration, l'exploration uniquement pour la recherche scientifique pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes et le rôle des grands fonds marins dans le système océanique et climatique, je vous donner un exemple : le projet de planeurs sous-marins français pour étudier le volcan sous-marin de Mayotte ou encore les campagnes en mer avec l'utilisation d'un drone, développé par une entreprise française et mise en oeuvre par l'Ifremer au milieu de l'Atlantique,

la France n'exploite pas dans ses eaux territoriales et nous sommes mobilisés pour convaincre les autres pays de s'engager dans cette voie de l'interdiction de l'exploitation en faisant tout cela sous l'égide de l'AFM, que nous aurons à transformer notamment sur la partie des financements, l'enjeu est bien évidemment d'être suffisamment de pays à défendre cette position pour que ce soit celles qui l'emporte, alors vous le voyez, les sujets de recherche sont nombreux, par la France et devront se faire en coordination avec les enjeux stratégiques de maîtrise des grands fonds marins de défense et de surveillance de nos territoires, c'est toute l'ambition de la stratégie du ministère des Armées qui accompagnent cette stratégie d'exploration des fonds marins, alors monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, cette ambition scientifique hé bien là et je sais que c'est une ambition collective partagée par le Sénat et à vous entendre, je fais le voeu ou en tout cas je suis convaincu que nous allons atteindre nos 2 objectifs : faire de la France un leader sur l'exploration des fonds marins avec un défi, celui de la connaissance scientifique pour ce que ce dernier espace inexplorée de la planète, soit mieux que nous, nos concitoyens et puis je terminerai par là, madame, monsieur le président, pardon sous-dotés des moyens pour accroître cette connaissance, l'émission que nous avons lancé permet aussi de tester les matériels français pour toujours être à la pointe en matière scientifique, je terminerai par une citation que je trouve très belle, en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles et donc continuons à porter son ambition maritime pour notre pays, merci de votre implication j'en vais vous dire, longue vie à la mère et la République élu. Merci, monsieur le Ministre. Merci, la parole est à monsieur Michel Canevet, président de la mission d'information exploration protection exploitation des fonds marins, quelle stratégie pour la France. Pour cinq minutes. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les différents orateurs des des groupes qui ont pu relayer le la vingtaine de recommandations que la mission a pu élaborer et puis donner bien entendu des éclairages particuliers sur un certain nombre d'aspects, je voudrais tout particulièrement remercier le rapporteur Téva Rohfritsch pour l'excellent travail qui a été menée remercie aussi l'équipe de collaborateurs menée par Catherine Forgeard qui a pu assister la mission pour que ce travail soit vraiment un travail efficace a audité, un certain nombre d'experts, plus de 60 experts et réalisé un gros travail, mais il faut dire que la dimension politique sur les fonds marins est absolument essentiel, il faut le rappeler et ceci bien sûr doit nous conduire à continuer à investir très largement dans les fonds marins parce que cela a été dit à de nombreuses reprises. Il y a pas grand chose de connu sur les grands formats, donc il faut qu'on continue l'exploration pour que la science puisse nous informer, de faire connaître tout ce qu'il y a de richesse dans les fonds marins et puis pour cela c'est clair, il faut des moyens, il faut des moyens, bien entendu, pour soutenir la recherche, il faut des moyens, cela a été dit tout à l'heure aussi pour le renouvellement de la flotte océanique, ce fut un des éléments qui ont permis à l'Ifremer, en particulier d'être particulièrement reconnu sur la scène internationale, au plan de la connaissance m'arrêter mais il importe que l'Ifremer puisse être dotée des outils du permettant de continuer à orienter les recherches et les mener bien entendu et j'intègre, bien entendu, la préoccupation de Philippe Folliot sur l'avenir du Nautile, qui est effectivement un outil extrêmement important, la France, c'est une ambition maritime, je suis heureux que Joël Guerriau est aussi à fermer la nécessaire ambition maritime de la Bretagne à 5 départements comme l'est actuellement la Normandie n'est-ce pas Jean Michel Houlgate il n'a pas de raison que nous soyons pas aussi bon que la Normandie mais surtout la Bretagne a de tout temps un lien historique très fort avec la mère et il importe que cela puisse continuer, alors vous l'avez dit, monsieur le Ministre des crédits ont été prévues dans le plan France 2030 322 millions d'euros, il faut effectivement que ces crédits puisse soutenir un certain nombre d'actions, alors pas seulement en subventionnant quelques projets, mais en accentuant je crois la la commande publique, nous l'avons constaté notamment par des par des rencontres avec les industriels, il importe que nous soyons actifs sur ce plan là, nous avons pu en Auvergne, en Norvège, particulièrement observé que, il y avait un soutien à la commande publique qui était opérant et qui ont permis à un certain nombre d'industriels, d'être aussi extrêmement efficace, il faut que la France puisse le faire aussi, et ça c'est important parce que nous ne sommes plus disons-le très clairement dans la science-fiction aujourd'hui on le voit, parce que bah notamment et il y a des autorisations qui ont été données pour l'exploitation à Nauru donc une filiale du Canadien TMC pour des explorations de Nobody nodules polymétalliques dans la zone de Clarion Clipperton, soyons clairs, donc tout ceci appelle notamment, vous l'avez dit à monsieur le ministre, à une consolidation de l'autorité internationale des fonds marins bien sûr pour un code minier qui soit efficace pour des moyens de contrôle qui soient accentuées pour un financement qui soient modifié et puis cela a été dit tout à l'heure aussi notamment par Joël Guerriau, la guerre des des fonds marins est aujourd'hui particulièrement importante, on l'a vu dans la mer Baltique, mais cela peut survenir aussi dans l'Atlantique dans la Méditerranée dans l'indo- Pacifique ou l'ado Océanie, il y a donc besoin de mener une protection extrêmement forte parce que nous avons des enjeux énergétiques des enjeux énergétiques des enjeux de télécommunications des enjeux de maintien de la biodiversité aussi qui sont essentiels dans ces régions, et donc il importe qu'là aussi, nous puissions nous préparer à ces enjeux futurs qui sont absolument nécessaires pour le 21 21ème alors je voudrais en concluant, vous dire que la question des des grands fonds marins est absolument importante dans notre pays parce qu'il y a des enjeux de souveraineté économique, cela a été dit de souveraineté, a dû Triel a dû Triel de souveraineté militaire, je viens d'en parler et puis aussi de souveraineté écologique, disons-le, ne l'oublions pas, et donc c'est un grand enjeu pour le 21 Itzhak, il faut que la France puisse y participer de toute sa place, il prend toute sa part, merci de votre attention et merci de la participation de tous à ce débat et aux propositions qui ont pu être formulées. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance mercredi 5 octobre à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement, la séance est levée.